la mission « Remboursements et dégrèvements » retrace les dépenses budgétaires résultant mécaniquement de l'application des dispositions fiscales prévoyant des dégrèvements d'impôts, des remboursements ou des restitutions de crédits d'impôt. Le caractère mécanique de ces dépenses implique que les crédits de la présente mission soient évaluatifs. En d'autres termes, ils ne constituent pas un plafond, contrairement à ceux des autres missions budgétaires. La mission est composée de deux programmes, l'un consacré aux remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, l'autre dédié aux mêmes opérations pour les impôts directs locaux, que je vous présenterai successivement, après avoir dit quelques mots de l'ensemble de la mission. Pour 2019, 135,7 milliards d'euros de crédits sont demandés au titre de la présente mission. Ce montant est en augmentation de 15 milliards d'euros environ par rapport à la loi de finances pour 2018. Il s'agit là d'un nouveau record pour cette mission. Cette augmentation très importante des crédits s'explique notamment, pour les impôts d'État, par la mise en oeuvre du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu et, pour les impôts locaux, par la deuxième tranche du dégrèvement de taxe d'habitation pour 80 % des Français et des Françaises. Au total, en 2019, les remboursements et dégrèvements devraient représenter un tiers environ des recettes fiscales brutes. Cette proportion, qui ne cesse d'augmenter après la parenthèse consécutive de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, traduit une politique fiscale qui repose de façon importante et croissante sur des mécanismes de réduction fiscale, lesquels grèvent en contrepartie les dépenses budgétaires et entravent les possibilités d'action de l'État. Le montant très important que représentent les remboursements et dégrèvements rendrait nécessaire une revue régulière et détaillée de leur pertinence. Absolument pertinence. Absolument ! Les remboursements et dégrèvements d'impôts d'État sont évalués à 115,8 milliards d'euros pour 2019. Ce montant est, lui aussi, en augmentation, de 7 milliards d'euros par rapport à l'année dernière, dans le prolongement de la hausse quasi ininterrompue de ces remboursements et dégrèvements depuis 2010. Un paramètre permet d'expliquer cette augmentation pour 2019 : l'entrée en vigueur du prélèvement à la source à compter du 1 janvier 2019. Le projet de loi de finances évalue les conséquences du prélèvement à la source à 11 milliards d'euros supplémentaires de remboursements et dégrèvements, en raison de l'acompte portant sur les crédits et réductions d'impôt de l'année précédente, qui sera versé en janvier 2019, et des restitutions d'excédents de crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement.

L'ensemble de l'effet budgétaire atteint quasiment 20 milliards d'euros en 2019. À partir de 2020, on pourra constater une diminution des remboursements et dégrèvements liés à ce dispositif, puisqu'il sera transformé en réduction de cotisations sociales employeurs l'année prochaine.

qu'inspire l'efficience de ce dispositif pour l'emploi, comme pour l'investissement ; j'observe que, sur ce sujet, un amendement sérieux a été déposé. J'en viens à la partie relative aux impôts locaux. Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux atteint le niveau record de 20 milliards d'euros, notamment du fait de la deuxième tranche du dégrèvement de taxe d'habitation pour 80 % des Françaises et des Français. Il continuera à croître en 2020, lorsque sera mise en oeuvre la troisième tranche du dégrèvement. Ainsi, dix ans à peine après la réforme de la taxe professionnelle, l'État redevient le premier contribuable local, dans la mesure où, en 2020, il prendrait en charge 22 % de la fiscalité économique et 37 % de la fiscalité « ménages

je souhaite profiter de l'examen de la présente mission pour évoquer l'avenir de la taxe d'habitation, qui devrait être supprimée d'ici à 2021, d'après le Premier ministre, et dont nous devrions débattre début 2019. Nous connaissons bien les limites de cette imposition, qui pèse parfois davantage sur les ménages modestes que sur les ménages aisés, sans qu'il soit possible de justifier de manière satisfaisante les écarts au sein d'une même commune. Cependant, je regrette que le Gouvernement choisisse de supprimer cette imposition plutôt que de la réformer pour qu'elle fonctionne de façon satisfaisante et juste. La taxe d'habitation représente un tiers des recettes fiscales du bloc local et plus de 20 % de ses recettes totales. Sa suppression déstabilisera les collectivités territoriales concernées en leur retirant un levier essentiel de leur action., c'est l'investissement local qui pourrait en pâtir, alors même qu'il représente 56 % de l'investissement public total et qu'il constitue un levier important pour la croissance. président. Pour ma part, je souhaite le maintien de la taxe d'habitation, associée à une mise en oeuvre rapide de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, qui résoudrait à mon avis une grande partie des difficultés posées par cette taxe.

Le montant global de la dette publique de l'ensemble des administrations publiques a temporairement dépassé le seuil symbolique des 100 % du PIB- ce chiffre est tout de même assez frappant ... La dette publique était à peine au-dessus du seuil des 60 points de PIB en 2007. Elle a augmenté de 40 points en dix ans

En d'autres termes, le gestionnaire d'infrastructure pourrait devenir, dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, une société anonyme à capitaux

il faudra faire très attention à la requalification de certaines dettes d'opérateurs de l'État en dettes publiques. Les pouvoirs publics peuvent être appelés à revoir les structures de gouvernance de ces opérateurs pour y diminuer la présence des représentants de l'État ou du Parlement. Les engagements hors bilan reflètent donc des niveaux de risque très divers et leur contrôle par le Parlement est variable, tendance faible ... Le troisième risque, c'est celui de la notation. À ce titre,

l'exercice auquel nous nous prêtons en ce début d'après-midi est pour le moins étrange. En effet, la présentation du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » s'opère de façon conventionnelle, avec un montant artificiel de crédits. Les impératifs de la LOLF sont aménagés afin de préserver la confidentialité des opérations de cession envisagées au cours de l'année suivante. Cette année, le montant conventionnel de crédits est multiplié par deux. choix artificiel est censé tenir compte des cessions envisagées par le Gouvernement et faisant l'objet de dispositions législatives dans le projet de loi dit « PACTE », que nous allons prochainement examiner. vous connaissez sans doute à grands traits le projet du Gouvernement. Il s'agit de céder 10 milliards d'euros de participations afin d'abonder un fonds pour l'innovation dite « de rupture », dont seuls les intérêts seront affectés à l'innovation. La dotation du fonds est donc non consomptible. Ce projet initial a été précisé dans le courant de l'année. Créé en janvier dernier, le fonds est placé auprès de l'EPIC Bpifrance. Il a reçu une dotation transitoire dans l'attente des cessions effectives d'Aéroports de Paris et de la Française des jeux, soit 1,6 milliard d'euros en numéraire, et des titres

Surtout, en août dernier, les modalités de placement de la dotation en numéraire du fonds ont été précisées. En pratique, les 10 milliards d'euros seront placés sur un compte ouvert auprès du Trésor, portant des intérêts annuels de 2,5 %. Compte tenu de ce taux, particulièrement avantageux dans le contexte actuel de taux faibles, je serais tenté de féliciter le Gouvernement pour ce rendement. La réalité est malheureusement plus sombre le rendement annuel du fonds de 250 millions d'euros sera retracé dans le budget général de l'État au titre du service de la dette. J'y vois tout simplement un tour de passe-passe. la dotation du fonds pour l'innovation viendra s'inscrire en déduction de la dette maastrichtienne. Par cet artifice, le Gouvernement affiche une réduction artificielle de l'endettement public. Le mécanisme du Gouvernement permet, en réalité, de contenir de 20 % le dérapage de l'endettement de l'État. Compte tenu de ce mécanisme, la commission des finances a adopté un amendement visant à réduire la contribution au désendettement assurée par le compte, dont le montant est doublé par rapport à l'an dernier. Il ne faudrait pas que l'État préempte les recettes des privatisations en empêchant le Parlement de donner son avis. Récapitulons les conséquences pour le budget général de cette opération : les dividendes tirés d'ADP et de la FDJ seront perdus, pour un montant moyen de 200 millions d'euros par an, tandis que les intérêts dus au titre de la dotation du fonds pour l'innovation s'élèveront à 250 millions d'euros par an. Or le Parlement ne sera nullement associé aux modalités du soutien à l'innovation qui sera apporté par le fonds.

La première nous est livrée par le Gouvernement lui-même : la dotation transitoire actuelle pourrait être prolongée, dans l'attente des retours des investissements consentis dans le cadre des PIA. Ces derniers sont estimés à près de 3 milliards d'euros d'ici à 2022, puis à 8 milliards d'euros d'ici à dix ans. C'est précisément le montant nécessaire pour compléter la dotation du fonds. La seconde consiste en une évolution du statut de l'Agence des participations de l'État. Actuellement, il s'agit sans doute du seul gestionnaire de participations qui ne bénéficie pas du produit des actifs qu'il gère. était dotée de la personnalité morale, elle pourrait percevoir ces dividendes. Elle serait liée à l'État par un contrat pluriannuel déterminant le montant du dividende annuel qu'elle serait tenue de lui verser. Cette évolution apporterait une solution aux deux difficultés principales actuellement constatées : d'une part, l'instabilité du montant annuel des dividendes perçus par l'État serait lissée ; d'autre part, l'information du Parlement ainsi que ses pouvoirs de contrôle seraient améliorés. L'équation insoluble entre l'information du Parlement et la confidentialité des opérations de l'État actionnaire, que le Gouvernement invoque pour justifier la mise à l'écart des deux assemblées, serait résolue.

Les PIA 1 et 2, d'un montant total de 47 milliards d'euros, font, eux, l'objet d'un suivi dans le cadre d'un jaune budgétaire. La loi de finances pour 2018 a inclus le PIA 3 dans le Grand Plan d'investissement et a doté la mission de ces premiers crédits de paiement à hauteur de 1,08 milliard d'euros. pour 2019 fait évoluer la maquette budgétaire en dotant la mission d'indicateurs de performance plus lisibles. Ces modifications, qui participent d'une meilleure information du Parlement, sont les bienvenues. Elles sont perfectibles : l'indicateur de performance des dispositifs de valorisation de la recherche pourrait inclure l'évolution du nombre de concessions de licences et de créations de start-up. En 2019, 1,05 milliard d'euros de crédits de paiement seulement sont inscrits. Ainsi, les crédits de paiement ouverts ne représentent que 21 % des 10 milliards d'euros d'autorisations L'effort budgétaire est repoussé vers la fin du quinquennat. Il est d'autant plus repoussé que les premiers crédits de paiement ouverts sont surtout ceux qui n'ont pas d'impact sur le déficit maastrichtien. Si la maquette n'évolue pas, certaines actions sont réorientées pour tenir compte du changement de politique depuis 2017, notamment dans le domaine de l'éducation. Cette mission étant jeune, nous pouvons encore l'aider à bien grandir. Sans prétention aucune, voici quelques pistes d'amélioration ou de vigilance. Tout d'abord, le décaissement des crédits de paiement sur plusieurs années induit des difficultés de gestion : premièrement, un dans le soutien à certains projets, qui provoque un décalage avec le rythme de vie des entreprises frilosité- les opérateurs attendent que les crédits de paiement soient disponibles pour finaliser les cahiers des charges ou commencent à financer les actions avec des aides d'un montant faible pilotage des projets par les opérateurs, non seulement par engagements, mais aussi par les décaissements, ce qui peut se traduire par une négociation projet par projet des priorités de paiements, avec, en conséquence, une hausse des coûts de traitement administratifs.

Ainsi, l'appel à manifestation d'intérêts lancé en mars 2018 pour l'action Créations expérimentales de sociétés universitaires et scientifiques n'a reçu aucune candidature. L'absence de crédits d'ingénierie pourrait expliquer cette inefficacité, les universités ou les écoles ne disposant pas, en interne, des compétences nécessaires à la constitution d'un dossier ou à la recherche d'investisseurs privés, qui doivent établir un socle minimum de financement du projet. De surcroît, l'articulation du PIA 3 avec le fonds pour l'innovation et l'industrie reste floue. Les 250 millions d'euros de dividendes annuels doivent se répartir entre 70 millions d'euros fléchés vers les start-up spécialisées dans les innovations de rupture et 150 millions d'euros destinés au financement des « grands défis de rupture deux grands défis seraient déjà identifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans le même temps, le projet annuel de performance du PIA 3 indique que l'action Programmes prioritaires de recherche devrait contribuer au financement du programme national pour l'intelligence artificielle, annoncé par le Président de la République le 29 mars 2018. Enfin, on observe un recours aux fonds du PIA pour financer les nouvelles politiques ou la relance industrielle territoriale. Ainsi, l'action Programmes prioritaires de recherche devrait contribuer au financement du programme de recherche consacré aux solutions alternatives aux produits phytosanitaires et à un programme de recherche dans le domaine du sport, dans la perspective des jeux Olympiques de Paris en 2024. Quant à l'action Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition, elle devrait participer au financement de la reconversion économique du site nucléaire de Fessenheim. Fessenheim. Le retard pris dans la publication de l'appel à projets sur le volet « territoires d'innovation de grande ambition » de la même action s'explique par la volonté du Gouvernement de recentrer l'action sur les « territoires d'industrie », dont le zonage doit être articulé à la carte des 222 villes du plan « Action coeur de ville Avant de céder la parole, je ne peux manquer d'évoquer la question de la rénovation du Grand Palais. D'après les informations communiquées, l'action Grands défis du programme 423 bénéficierait avant 2021 d'un redéploiement de 200 millions d'euros de subventions pour contribuer au financement de la rénovation de ce monument parisien. Le plan de financement de la rénovation présenté par nos deux rapporteurs spéciaux du budget de la culture confirme cette hypothèse. À mon sens, on ne peut que regretter un tel détournement de l'esprit du PIA. même si nous sommes loin de l'esprit du rapport remis par Jean Pisani-Ferry en septembre 2017, je vous recommande d'adopter les crédits de la mission. Nous nous retrouverons l'année prochaine, pour voir si la situation a évolué dans un sens meilleur.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, sur le rapport de notre collègue Alain Chatillon, empêché, la commission des affaires économiques a regretté une nouvelle fois la présentation « conventionnelle des recettes et des dépenses du compte, même si elle prend en considération pour 2019 des opérations de cession conditionnées à l'adoption du projet de loi PACTE, à savoir les cessions de titres d'Aéroports de Paris et de la Française des jeux. l'allocation du produit de ces cessions suscite des interrogations, avec, au premier chef, l'abondement du fonds pour l'innovation et l'industrie. D'une part, sur le principe, on peine toujours à comprendre l'intérêt financier de cette opération : il s'agit de céder des titres dont le rendement est de 3,5 % par an pour les placer à un taux inférieur à 2,5 %. Il serait plus judicieux financièrement, et plus simple en pratique, d'affecter directement une partie des dividendes dégagés par le portefeuille de l'État au financement de l'innovation. La constitution provisoire du fonds depuis janvier 2018, par apport de titres d'EDF et de Thales, a d'ailleurs montré que le portefeuille de l'État était parfaitement à même d'assurer un rendement semblable. D'autre part, cette cession risque de réduire les capacités futures d'intervention de l'État. En effet, c'est le portefeuille de ses participations qui lui a donné les moyens destinés à restructurer la filière nucléaire française en 2016 ou à recapitaliser des entreprises stratégiques, comme PSA en 2014. L'État doit donc conserver des marges de manoeuvre et éviter de vendre les bijoux de famille. Plus généralement, la commission souhaite appeler l'attention du Sénat sur le déficit d'information du Parlement, quant à la gestion par l'État de ses participations dans les entreprises. d'abord, un fort décalage ne peut être exclu entre les prévisions conventionnelles affichées par le CAS et la réalité de l'exécution du compte. Ensuite, le Parlement n'est pas mis en mesure de participer effectivement à la définition de la stratégie de l'État actionnaire. Nous le déplorons. Il faut donc trouver les moyens d'associer en amont le Parlement aux décisions. Il faut que le Gouvernement informe et consulte périodiquement les commissions permanentes compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale, au sujet de la stratégie de cession ou d'acquisition d'actifs qu'elle entend mener, dans le respect de la confidentialité qui s'attache aux informations relatives aux décisions de cession ou d'achat d'actifs. On peut penser à des échanges en commission restreinte ou à huis clos, le cas échéant, avec un engagement à respecter le caractère confidentiel des données transmises. Le projet de loi PACTE fournira le support législatif idoine.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote.

ainsi que les comptes d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » et « Participation de la France au désendettement de la Grèce », dont le contenu est pour l'essentiel la conséquence de la politique menée au cours des dernières années, voire des dernières décennies. Ces missions ne suscitent pas de critiques majeures de la part des élus du RDSE. Nous approuverons donc les crédits dont il s'agit, à moins qu'ils ne soient profondément modifiés par certains amendements. Ils méritent toutefois quelques remarques et suscitent un certain nombre d'interrogations. Les engagements financiers de l'État relèvent essentiellement de la charge de la dette, qui représente la quasi-totalité des crédits. Elle est relativement stable depuis plusieurs années, à un peu plus de 42 milliards d'euros, soit une légère hausse de 1,02 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. Cette stabilisation a pour origine des taux d'intérêt extrêmement bas, qui ont néanmoins commencé à légèrement remonter cette année. L'encours de la dette continue d'augmenter. Il devrait atteindre 98,7 % du PIB en 2019, alors que la majorité des États de la zone euro connaissent désormais une trajectoire inverse, à la baisse. Le besoin de financement progresse également en raison de cette majoration et de l'arrivée à échéance de certains titres émis lors de la crise financière de 2008-2009. Cette situation fait peser sur nos finances publiques des risques, dont le plus important est la remontée des taux d'intérêt, qui commence à se matérialiser. Il est donc nécessaire de poursuivre et d'accentuer les efforts pour engager un réel désendettement, et non plus seulement une contribution au remboursement de la dette, comme c'est le cas aujourd'hui. La mission « Investissements d'avenir », qui trouve ses origines dans les travaux d'une commission présidée, il y a une décennie, par Alain Juppé et Michel Rocard, illustre la volonté des gouvernements successifs de soutenir de manière dynamique et sélective les actions porteuses d'avenir pour notre économie. Elle souligne en même temps la difficulté de mettre en oeuvre rapidement les mesures d'incitation ou d'accompagnement choisies dans différents programmes. Les trois programmes d'investissements d'avenir ont été réunis l'an dernier au sein d'un Grand Plan d'investissement de 57 milliards d'euros. de loi de finances pour 2019 par l'inscription de 1,05 milliard d'euros en crédits de paiements. Ce montant est relativement modeste et ne paraît pas être à la hauteur de l'ambition affichée de doter notre pays d'une économie performante. On ne peut pas réduire une logique de projet à une stricte logique budgétaire, même si, en agissant ainsi, le Gouvernement est dans son rôle. La mission « Remboursements et dégrèvements », qui recouvre 115,8 milliards d'euros de crédits en 2019, est en hausse de 7 milliards d'euros par rapport à 2018, soit une hausse un peu moins forte que l'an dernier, mais tout de même importante, qui résulte, notamment, de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, du poids persistant du CICE, ainsi que de la censure par le Conseil constitutionnel du mode de calcul de la CVAE.

Enfin, j'évoquerai les comptes d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » et « Participation au désendettement de la Grèce ». Le premier est le support budgétaire de l'État actionnaire. Sa particularité est de présenter une programmation conventionnellement à l'équilibre afin de préserver la confidentialité des opérations de cession ou d'acquisition à venir.

Le montant des crédits dédiés à la charge de la dette représente le poids du passé, qui obère nos politiques publiques aujourd'hui et pèsera, demain, sur les épaules de nos enfants. À l'inverse, les investissements d'avenir constituent un effort salutaire, mais bien modeste en comparaison, pour préparer le futur de notre économie et de notre société. Je commencerai par évoquer le poids du passé : la dette. Le programme 117 de la mission « Engagements financiers de l'État », qui représente la quasi-totalité des crédits de la mission, contient la charge d'intérêts de notre dette souveraine. de loi de finances pour 2019 un montant de 42,47 milliards d'euros, en croissance de 1,7 % par rapport à 2018. C'est six fois le budget de la justice ou encore 10 milliards d'euros de plus que le budget de la défense. On mesure ainsi le gaspillage de ressources auquel nous consentons chaque année. Malgré les efforts du Gouvernement, la dette française continue donc de s'accroître inexorablement, alimentée par des déficits qui ne se résorbent que trop lentement. Nous l'avons rappelé lors de la discussion générale, la réforme de l'État menée par le Gouvernement, notamment dans le cadre du Comité Action publique 2022, va dans le bon sens. Elle reste néanmoins très insuffisante pour réduire vigoureusement la dépense publique et combler notre retard sur d'autres pays européens, en particulier sur l'Allemagne. Notre trajectoire de désendettement, par exemple, est nettement en deçà de celle de nos voisins

Ce différentiel d'endettement avec l'Allemagne en 2022 sera sans précédent dans l'histoire récente de l'Europe. Il augure une perte d'influence durable de la France face à des partenaires disposant de marges de manoeuvre plus importantes pour agir et, par conséquent, pour décider. Si nous ne parvenons pas à maîtriser plus sérieusement les dépenses de l'État, qui ont progressé de 20 % entre 2007 et 2016 ; si nous ne parvenons pas à résorber nos déficits effectifs et structurels de façon plus volontaire ; et si, enfin et en conséquence, nous ne parvenons pas à diminuer le stock de notre dette de manière forte, c'est bien notre stature politique en Europe et dans le monde qui en pâtira. Il ne s'agit pas ici que de chiffres, mais il s'agit bel et bien de notre capacité à agir.

J'en viens à un aspect qui nous rend plus optimistes : les crédits dédiés à la mission « Investissements d'avenir ». Leur objectif est d'augmenter la croissance potentielle de la France, en misant sur l'économie de l'intelligence, sur l'innovation et sur la recherche. Leur montée en puissance, tant quantitative que qualitative, doit être saluée, mais nous nous interrogeons sur leur articulation avec le fonds pour l'innovation et l'industrie prévu par le Gouvernement. La gamme des outils mobilisés nous semble également pertinente. Je rends aux travaux de notre collègue Christine Lavarde sur le dispositif des avances remboursables, qui montrent que cet outil est très utile, notamment pour les PME. Leur usage pourrait être davantage développé. Le groupe Les Indépendants-République et Territoires votera les crédits de ces missions, en espérant avoir plus de raisons encore de le faire l'année prochaine.

ces prévisions sont entachées d'un certain nombre d'aléas, parmi lesquels les tensions commerciales avec les États-Unis et le retour de la volatilité sur les marchés financiers. Dans ce contexte, et non sans prudence, le Gouvernement a choisi une hypothèse de croissance de 1,7 % pour 2019, comme, d'ailleurs, pour les budgets à venir jusqu'en 2022. En 2019, l'encours de la dette négociable de l'État va poursuivre sa progression, avec une augmentation de 84 milliards d'euros par rapport à 2018, pour atteindre 1 845 milliards d'euros, soit deux fois le niveau de 2007. Cela résulte également d'une normalisation des conditions de financement de l'État, avec une remontée progressive des taux d'intérêt ainsi qu'une reprise de l'inflation. La durée de vie moyenne de la dette négociable de l'État continue de s'allonger et s'établit à 7 ans et 325 jours à l'automne 2018,

un mot sur un nouveau produit de la dette : l'OAT verte. Émise par la France depuis janvier 2017 pour un montant initial de 7 milliards d'euros, mais dont l'encours atteint aujourd'hui presque 15 milliards d'euros. du Trésor verte permet de financer quatre objectifs : la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité ou encore la lutte contre la pollution. L'OAT verte est un instrument intéressant qui permet de rendre plus transparentes les dépenses environnementales de l'État, notamment en matière de transition énergétique. Je souhaite également dire un mot des investissements d'avenir, qui font désormais partie du Grand Plan d'investissement d'un montant de 57 milliards d'euros sur le quinquennat et dont je rappelle les quatre points cardinaux : accélération de la transition écologique, développement d'une société de compétences, ancrage de la compétitivité sur l'innovation et construction de l'État de l'âge numérique.

j'appelle votre attention sur le rapport de la Cour des comptes publié en mars 2018, qui nous invite à regarder les résultats de ce plan. La Cour recommande notamment de « resserrer le périmètre des outils du PIA » pour « améliorer les conditions de valorisation de la recherche publique.

Le projet de loi sur les finances locales, qui sera, selon toute vraisemblance, présenté au premier semestre, permettra de débattre du bouclage financier total de cette exonération.

Participations financières de l'État » soit fixé de manière conventionnelle à 5 milliards d'euros. Pour l'année 2019, le projet de loi de finances double la prévision de recettes en la portant à 10 milliards d'euros. Cette hausse prévisionnelle découle des privatisations envisagées l'année prochaine par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi PACTE, qui sera bientôt examiné au Sénat. L'État entend ainsi se séparer d'Aéroports de Paris, de la Française des jeux et d'Engie.

un non-sens économique, parce que le Gouvernement estime lui-même que ce fonds pour l'innovation ne serait doté chaque année que de 250 millions d'euros, distribués sous forme de prêts ou d'avances remboursables. Cette somme correspond aux dividendes issus du placement du capital obtenu par la cession des actifs en question.

avec une progression moyenne de 10 % du résultat net observé lors des dix dernières années, on estime que, d'ici à cinq ans, les seuls dividendes perçus d'ADP pourraient financer la

réalisés pour l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, qui permettront d'augmenter sa capacité de 10 millions de voyageurs. Il est également question d'améliorer sa desserte grâce à l'efficience de sa plateforme multimodale et de créer un quartier d'affaires international dans le cadre du projet « Coeur d'Orly Pourquoi nous séparer d'infrastructures aussi stratégiques ? Pourquoi perdre la maîtrise de cette entreprise, alors qu'il est possible de flécher, tout simplement, la totalité des dividendes perçus d'ADP vers ce fonds pour l'innovation Autrement dit, pourquoi choisir une privatisation plutôt qu'une optimisation des dividendes actuellement perçus, au regard de leur produit ? Ce sont des questions essentielles qui sont posées au Gouvernement, lequel, à l'heure actuelle, ne nous a toujours pas démontré l'efficacité d'une telle opération. Bien au contraire ! Dois-je rappeler comment ce gouvernement a décidé de céder

Je n'ai pas encore évoqué la privatisation de la Française des jeux, qui laissera l'État gérer et supporter seul les dépenses sociales liées aux addictions et au surendettement sans même percevoir des dividendes. Les plus grandes craintes ont également été exprimées à l'Assemblée nationale quant à un désengagement de la Française des jeux du financement du sport, un domaine déjà fortement amputé dans le projet de loi de finances pour Permettez-moi de faire ici le lien avec l'incohérence et le non-sens stratégique que j'évoquais au début de mon propos. L'année dernière, j'avais déjà souligné le danger de perdre la main sur des entreprises stratégiques pour notre pays. Je le redis cette année avec force : ces cessions risquent de considérablement diminuer les capacités

nous persistons et nous signons : ce fonds pour l'innovation et l'industrie n'a pas remplacé et ne remplacera jamais la volonté politique d'un État stratège pour soutenir à tout moment nos entreprises nationales,

nous nous séparons de bijoux industriels, de grandes entreprises nationales. Ce n'est certainement pas la bonne méthode pour faire face à la mondialisation qui est devant nous ! La parole est

Malgré la volonté des gouvernements successifs, nous constatons malheureusement que la dette publique poursuit depuis longtemps son inquiétante envolée : elle se situe aujourd'hui à près de 100 % du PIB.

le défi de l'endettement public n'est pas nouveau, mais il se fait de plus en plus pressant et redoutable. Sur ce sujet, nous faut, ensemble, faire preuve de la plus grande responsabilité ; nous le devons aux générations à venir. Nous ne pouvons plus continuer à réclamer sans cesse l'allégement des prélèvements obligatoires et la réduction de la dépense publique sans avoir collectivement le courage de définir précisément les dépenses qu'il convient de réduire. Monsieur le secrétaire d'État, il me semble urgent de définir une stratégie à court, moyen et long terme pour diminuer durablement notre endettement en agissant sur deux leviers un plan de réduction de la dépense publique, dont je m'empresse de dire qu'il ne devra pas pénaliser les plus démunis de nos concitoyens ni accroître la fracture territoriale, et une lutte plus offensive et plus efficace contre la fraude fiscale, dont on sait qu'elle représente chaque année l'équivalent de notre déficit. déficit. La mission « Investissements d'avenir » procède à la mise en oeuvre d'un troisième programme d'investissements d'avenir. La programmation pour la période triennale 2018-2020 est scrupuleusement respectée, et nous tenons à le saluer

Il faudra toutefois veiller à ce que la redéfinition de certaines actions et priorités ne menace pas les projets qui, depuis l'origine, sont au coeur des enjeux du PIA 3. Enfin, la mission « Remboursements et dégrèvements » retrace les dépenses budgétaires résultant mécaniquement de l'application des dispositions fiscales : dégrèvements d'impôts, remboursements, restitutions de crédits d'impôt, compensations.

2019, sert à accompagner les ménages dans cette transition. Vous avez, à juste titre, mis en place un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, dont le coût est évalué à 6,9 milliards d'euros et qui vise à neutraliser le passage au prélèvement à la source.

Nous saluons les précautions prises par le Gouvernement pour que cette année de transition se passe le mieux possible pour l'ensemble des ménages, en particulier pour les plus vulnérables, auxquels sont accordés des avantages de trésorerie significatifs. La seconde spécificité de cette année tient aux remboursements et dégrèvements d'impôts locaux, en hausse de 3,8 milliards d'euros. Cela correspond simplement à la deuxième année de mise en application de la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages. Le mécanisme de dégrèvement par lequel l'État se substitue au contribuable dans le paiement de la taxe d'habitation permettra aux collectivités locales de conserver l'intégralité de leurs recettes ; nous nous réjouissons de ce choix qui les préserve. Lors de l'examen, Lors de l'examen, au printemps 2019, du projet de loi spécifiquement dédié à la refonte de la fiscalité et des finances locales, nous aurons l'occasion de revenir sur les mécanismes de compensation qui devront être mis en oeuvre à l'horizon de 2020, lorsque la taxe d'habitation sera

Elle comportait alors une enveloppe de 10 milliards d'euros au titre des autorisations d'engagement visant à mettre en oeuvre le troisième programme d'investissements d'avenir. Toutefois, aucun crédit de paiement n'était inscrit. Qu'en est-il du projet de loi de finances pour 2019 ? Le PIA 3, qui s'était vu attribuer 1,08 milliard d'euros en crédits de paiement en 2018, continue sur sa lancée et bénéficie de 1,05 milliard d'euros. Le projet de budget pour 2019 est, par conséquent, conforme à la programmation triennale 2018-2020 annoncée il y a un an, qui prévoyait 4 milliards d'euros sur les trois années.

qu'il s'agisse de la répartition des autorisations d'engagement inscrites ou des actions et des programmes qui la constituent. Permettez-moi néanmoins de rejoindre les propos de Mme le rapporteur spécial et d'appeler votre attention sur les conséquences que pourrait engendrer le choix du Gouvernement de lier les décaissements des crédits du PIA 3 aux contraintes budgétaires. Il me semble en effet important de garder en tête que le choix d'un décaissement progressif des crédits de paiement ne sera pas sans conséquence sur le bon déroulement du PIA, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, force est de constater que l'ouverture progressive des crédits de paiement risque de ralentir la mise en oeuvre des actions. Dans son rapport, notre collègue rapporteur spécial évoquait à ce titre deux conséquences du décalage du décalage temporel entre décaissement des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, évoquées par les opérateurs à l'occasion des auditions : d'une part, le problème du, qui se qui se pose dans le soutien à certains projets, provoque un décalage avec le rythme de vie des entreprises et expose au risque d'à-coups dans la mise en oeuvre du PIA ; d'autre les opérateurs reconnaissent qu'une certaine frilosité les conduit à attendre que les crédits soient disponibles avant de finaliser le cahier des charges et de lancer l'appel à projets ou de commencer le financement des actions avec des « tickets » de taille inférieure. Ensuite, le fait que les crédits de paiement ne soient pas intégralement ouverts et versés aux opérateurs conduit à une gestion différente des actions par ces derniers, qui opèrent davantage sous contrainte. Je pense notamment au suivi informatique, qui nécessite dès lors un pilotage non plus seulement par les engagements, mais également par les décaissements, afin de veiller à ce que les décaissements de l'année soient inférieurs ou égaux aux plafonds de crédits de paiement imposés. je conclurai mes propos en rappelant la nécessité de veiller à ne pas multiplier les aides à l'innovation, ce qui revient finalement à saupoudrer l'argent public ici et là. Il me semble incontestable que doublonner les aides à l'innovation ne conduirait à rien, si ce n'est à déboussoler ou désorienter les porteurs de projets. je citerai plus spécifiquement le récent fonds pour l'innovation et l'industrie, initiative du GPI, et dont l'articulation avec le PIA 3 apparaît fragile. Dans cette optique, au-delà de la proximité sémantique entre les « grands défis » du PIA 3 et ceux du je me dois de relever la proximité des projets que financerait le fonds pour l'innovation et l'industrie avec les actions soutenues dans le cadre du PIA 3. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ne disposant que de cinq minutes, je concentrerai mes propos sur deux aspects. Les dégrèvements, à qui profitent-ils ? Pour 101 milliards d'euros, aux entreprises ! Ça alors ! Je souhaite évoquer le rapport d'étape de France Stratégie sur la mise en oeuvre du CICE. l'emploi, c'est 20 milliards d'euros par an de cadeaux aux entreprises- 99,3 milliards depuis 2013 ! Selon ce rapport, « on sait peu de choses sur la nature des emplois créés ou sauvegardés », « les conséquences à moyen et long terme sur l'appareil productif sont largement inconnues ». Enfin, « on ne dispose d'aucune étude sur leurs effets sur la formation, les investissements, l'innovation, la montée en gamme de l'économie française et sur la croissance

Le CICE a donc été une ristourne fiscale et un dispositif de baisse du coût du travail. Vous me direz que le CICE ne vise pas que l'emploi. le rapport souligne « qu'il y a une absence d'effet ou un effet très limité, et même nul, du CICE en matière d'exportations, d'investissements, de salaires, de taux de marge, de recherche-développement, voire de création d'emploi

Et c'est avec nos impôts, monsieur le secrétaire d'État, qu'on licencie aujourd'hui en France ! Si on combine les aides de l'État, les exonérations de cotisations sociales, les aides régionales et européennes, on se retrouve avec près de 6 000 dispositifs, comme le montre bien le site, destiné aux futurs entrepreneurs. On se rend alors compte que le capital coûte près de 200 milliards d'euros par an. Et pourtant,

Après la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, après la, après la suppression de l', vous décidez de poursuivre avec le CICE, et même de le pérenniser sous forme d'allégements de cotisations patronales. Et comme on peut le faire à la Française des jeux, vous doublez la mise : 40 milliards d'euros, alors que, dans le même temps, les dotations des autres missions du budget de l'État sont affaiblies. Pour finir, je voudrais vous parler de la cession des titres détenus par l'État, en me concentrant sur ADP. Comme le souligne très justement le rapporteur spécial, la valorisation boursière d'ADP a été multipliée par quatre en dix ans. Ce groupe a versé à l'État un dividende de 132 millions d'euros en 2017. Je sais que nous avons des débats entre nous sur les privatisations, mais quand on confie au secteur privé un monopole naturel comme celui d'ADP, c'est un peu comme s'il obtenait le billet gagnant du loto chaque semaine. Rappelons-nous, chers collègues, le scandale de la privatisation des autoroutes.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs,

Nous avons parlé de ce dont nous héritons, le patrimoine de l'État, de ce que nous construisons, le plan d'investissements d'avenir, et puis de cette dette, qui était là, qui sera là, et à laquelle il faut donner du sens. les participations financières de l'État, il s'agit d'abord de respecter les engagements pris. Il s'agit ensuite de financer l'innovation et de contribuer au désendettement.

pouvant résulter des cessions permises par la loi PACTE, ainsi que de l'engagement de consacrer principalement ces recettes au fonds pour l'innovation et l'industrie et au désendettement de l'État. Vous avez parlé du passé et de la nécessaire préservation des intérêts patrimoniaux de l'État. De manière constante, tous les gouvernements ont fait le choix de retenir un montant notionnel de prévisions de recettes et de dépenses afin de ne pas donner de signaux aux marchés. Le Gouvernement est soumis à une double obligation : celle d'information et de transparence à l'égard du Parlement et celle de gérer au mieux les deniers publics face aux marchés,

Enfin, nous veillons à l'augmentation de la valeur des participations financières de l'État. Depuis le début de cette année, le portefeuille coté de l'État poursuit sa très bonne performance. Il est important de le souligner. En ce qui concerne le programme d'investissements d'avenir, comme vous le savez, le Gouvernement s'est engagé dans une politique d'investissements volontariste pour accompagner les réformes structurelles que nous portons et répondre aux défis majeurs de la France. C'est le sens du Grand Plan d'investissement lancé par le Premier ministre, le 25 septembre dernier, et qui va se déployer tout au long du quinquennat. Le troisième volet du programme d'investissements d'avenir est une composante pleine et entière de ce GPI. Il contribue directement à ses champs d'intervention prioritaires : accélérer la transition écologique, édifier une société de compétences, ancrer la compétitivité sur l'innovation, construire l'État de l'âge numérique. Avec le PIA 3 et ses 10 milliards d'euros, actés par la loi de finances pour 2017, l'État s'est donné les moyens de transformer profondément le tissu économique français. Ainsi, le PIA 3 n'est pas structuré par secteur, mais de l'amont à l'aval, de l'enseignement et la recherche jusqu'à l'innovation et le développement des entreprises, autour de deux vecteurs de transformation : la transition à l'heure d'un monde numérique et l'impératif de développement durable. Sur la nature des crédits, entre fonds propres et avances remboursables, le PIA 3 fait une large place aux fonds propres, avec près de 4 milliards d'euros, afin de valoriser économiquement l'effort exceptionnel consenti pour la recherche et l'innovation des PIA 1 et 2, en partageant mieux les risques avec les entreprises et donc également les perspectives de rentabilité en cas de succès.

1 milliard d'euros en crédits de paiement seront ouverts en 2019 afin de concrétiser ces ambitions, conformément à la trajectoire triennale, ce qui correspond à une montée en charge progressive des décaissements directement liée à la programmation et aux mécanismes des différents dispositifs.

fonds marque notre volonté d'amplifier l'effort en faveur de l'innovation de rupture en ciblant prioritairement les entreprises à très forte intensité technologique, en assumant une prise de risque plus grande, notamment s'agissant des grands défis que nous avons annoncés, avec le ministre de l'économie et la ministre de la recherche.

grâce à une réduction du poids de la dépense publique de plus de 3 points et à une diminution des prélèvements obligatoires de 1 point, ainsi qu'une baisse du ratio de dette publique d'au moins 5 points à l'horizon du quinquennat à l'aide de réformes structurantes et volontaires que vous avez Je tiens à vous répéter notre détermination à redresser durablement les finances publiques françaises, un redressement allant de pair avec les réformes structurelles que nous menons pour rendre la France toujours plus attractive. je vous rappelle que les crédits de cette mission comportent également les appels en garantie liés aux dispositifs de garantie à l'export que nous avons profondément modernisés et renforcés, notamment avec la réforme de l'assurance prospection, dont le plein effet budgétaire ne se fera sentir qu'en 2020, ainsi que ceux liés au soutien à l'accession à la propriété dont les encours augmentent, mais la sinistralité reste très faible. Vous l'aurez compris, c'était à la fois une réflexion sur le passé et sur le présent. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission

ce dont je doute

ces cinq dernières années, le cours de son action est passé de 74 à 193 euros. ADP représente près de 5 % du PIB régional, 1,4 % du PIB national et génère 8 % des emplois régionaux et 2 % de l'emploi national. Il s'agit donc d'un actif particulièrement important pour l'État, lequel a perçu plus de 1,1 milliard d'euros de dividendes en dix ans. De plus, en 2017, ADP a été le point d'entrée sur le territoire de plus de 100 millions d'individus.

Nous ne développerons pas ici les enjeux en termes d'investissements, de sécurité des infrastructures et d'unité du système aéroportuaire. Nous ne développerons pas non plus la question de l'avenir du Grand Paris, dans lequel ADP occupe une place centrale, sans parler de la maîtrise du foncier, avec le risque d'une spéculation encore plus effrénée, nocive pour les communes avoisinantes et leurs habitants. Ainsi, alors même que la décision de privatiser les aéroports de Toulouse et de Nice est aujourd'hui largement critiquée, vous maintenez le cap, même s'il vous mène droit dans le mur. En cédant cette entreprise, vous agissez contre les intérêts de notre pays. Et pour quels motifs ? Vous évoquez un fonds d'innovation de rupture ayant vocation à moderniser et à enrichir l'économie nationale et qui sera donc financé par la cession d'un groupe rapportant, chaque année, des dividendes importants à l'État.

qui n'est pas rien. La cession envisagée privera donc l'État de ressources financières importantes, alors même que la Française des jeux n'aura pas besoin d'investissements importants. De plus, ce désengagement de l'État dans la Française des jeux vient tourner le dos à notre tradition républicaine de régulation des jeux d'argent.

un amendement qui vise à abaisser les prélèvements de l'État en matière de désendettement, préemptant ainsi, si j'ose dire, les recettes futures de privatisation.

compte tenu des taux faibles auxquels l'État se finance actuellement sur les marchés financiers, il ne paraît pas souhaitable de multiplier par deux

de deux risques identifiés pour 2019 : d'une part, le caractère improbable de l'encaissement dès 2019 du produit tiré de la cession des titres de participation de l'État dans la Française des jeux et, d'autre part, le risque résultant d'un solde cumulé du compte s'établissant à un niveau très faible pour la capacité de réaction de l'État actionnaire. En effet, en cas de survenance d'un risque systémique imprévu et à défaut de réserves suffisantes sur le compte, un versement du budget général serait nécessaire, ce qui assujettirait l'État actionnaire aux contraintes inhérentes à la gestion budgétaire annuelle.

Les cessions de participations ne sont pas motivées par des besoins de trésorerie, je l'ai rappelé précédemment. Le Gouvernement a défini une trajectoire budgétaire pour le quinquennat, et il la respectera. Il faut que l'État soit plus sélectif dans l'utilisation des deniers publics et limite l'immobilisation

s'agit d'utiliser l'argent public pour investir dans les technologies de demain et réduire l'endettement, parce que la dette est un poison lent et puissant pour l'économie française. La logique du dispositif qui a été retenu est de céder des participations, plutôt que de les gérer passivement, et d'investir le produit des cessions dans un fonds dont le rendement financera durablement et de façon stable les innovations de rupture. Ce fonds a vocation à s'inscrire dans une durée longue, comme un outil de long terme pour le financement de ces innovations.

nous avons été un certain nombre à vouloir restaurer la pratique de l'évaluation de nos politiques publiques. Or, ici, nous ne

Le meilleur moment pour privatiser une entreprise et pour défendre au mieux les deniers de l'État et, donc, de nos concitoyens, c'est quand elle est en bonne santé

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

destiné en particulier à flécher des financements pour soutenir la transition numérique de ces entreprises. Les entreprises artisanales rencontrent souvent des difficultés pour financer leur développement, en particulier leur transformation numérique. En effet, les outils financiers existants exigent des seuils de chiffres d'affaires trop élevés pour rendre ces entreprises éligibles aux dispositifs en vigueur. Rappelons que 41 % des artisans seulement ont un site web, 15 % procèdent à de la vente en ligne et 25 % utilisent les réseaux sociaux. Il importe donc de permettre aux entreprises artisanales de s'inscrire dans le Grand Plan d'investissement. À cette fin, l'amendement vise à flécher 50 millions d'euros de crédits de paiement de l'action n° 02, Accompagnement et transformation des filières, du programme 423, « Accélération de la modernisation des entreprises vers le financement d'un nouveau programme dédié au fonds d'innovation et de développement des entreprises artisanales, dont les modalités de mise en oeuvre seront fixées par décret.

qui vise à réaliser des investissements, un fonds géré par Bpifrance, dans des sociétés de projets créées par plusieurs entreprises d'une même filière dans le but de favoriser la transformation de ladite filière. Des crédits pourraient notamment être consacrés,

M. Emmanuel Capus. Favoriser les PME de croissance est une cause nationale pour l'économie et l'emploi. Si l'économie ne repart pas en France, c'est en particulier à cause d'un déficit d'exportations, lié à un problème chronique d'offre de la part d'entreprises qui ne sont pas assez compétitives, notamment dans l'industrie. Sur les neuf premiers mois de l'année 2018- je l'ai dit lors de la discussion générale -, le déficit cumulé de la France a ainsi atteint 48,2 milliards d'euros, ce qui est une cause de faiblesse et de dépendance structurelle pour notre économie.

passe par l'internationalisation de nos ETI et de nos PME, qui n'ont pas la même facilité à exporter que leurs homologues allemandes. Dans le cadre des investissements d'avenir, il importe ainsi de leur apporter un soutien fort dans cette démarche-

Cela ne signifie pas que, programme par programme, il n'y ait aucun point positif- j'y reviendrai -, mais ce budget traduit d'abord une politique que nous devons apprécier dans son ensemble et, avant tout, à l'aune de ses résultats ; or nous en constatons les premiers effets en matière de logement. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, monsieur le ministre. L'an dernier, ici même, sur toutes les travées, et en juillet encore, lors de l'examen de la loi ÉLAN, la bien mal nommée, nous avons dit et répété que vos choix politiques et budgétaires auraient des conséquences dramatiques. Nous y sommes Les derniers chiffres montrent une chute inquiétante des réservations pour la promotion privée, et le nombre de logements sociaux financés repassera probablement cette année sous le seuil des 100 000. L'an dernier, et à l'été encore, vous vous vouliez rassurant. Les fameuses mesures de compensations de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la loi ÉLAN, qui mettra du temps à produire ses effets, allaient permettre aux acteurs du secteur d'encaisser le choc budgétaire. Grave erreur ! La reconnaîtrez-vous enfin et en tirerez-vous les conséquences ? Votre politique a un but : réaliser des économies budgétaires. Elles sont là. Mais à quel prix ? Moins de logements dès cette année, moins d'emplois demain, mais aussi moins de rentrées sociales et fiscales pour l'État. C'est donc dans ce contexte difficile que nous examinons les crédits de la mission. par la LOLF, il ne nous est pas possible de modifier le cours que vous avez donné aux choses. Mais nous voulons, une fois encore, tirer le signal d'alarme. La mission est dotée cette année de 16,1 milliards d'euros de crédits de paiement, mais, vous le savez, le programme 109 en porte l'essentiel,

la transition énergétique. S'agissant du programme 177, « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », il est à noter que la gestion des centres d'hébergement d'urgence dédiés aux migrants d'Île-de-France est enfin transférée à la mission « Immigration et asile ». Voilà un point de clarification budgétaire bienvenu ! Abstraction faite de cette mesure de périmètre, les crédits de paiement sont en hausse de 43 millions

sociale, sont réduits de 14 millions d'euros, alors même que le plan Logement d'abord, lancé à l'automne 2017, tarde vraiment à produire des résultats. Cependant, j'interprète ce chiffre non pas comme une réduction du nombre de places offertes, mais, en partie, comme le résultat de la poursuite de la convergence tarifaire entre structures.

budgétaire : la sous-revalorisation des aides- 0,3 % -par rapport à l'inflation- 1,6 % -et la prise en compte des revenus contemporains des allocataires, qui impactera d'abord, soyons-en conscients, les jeunes qui entrent sur le marché du travail, qui se verront dès lors réduire ou couper l'APL bien plus rapidement qu'avant. Se pose également la question du rendement de cette mesure : annoncée à hauteur de 1,2 milliard d'euros en année pleine, elle ne pourra finalement être mise en oeuvre avant juillet. Pourtant, le Gouvernement retient toujours un gain de 900 millions d'euros en 2019. Cela mérite quelques explications. Soulignons enfin le risque pointé par la CAF, qui, si elle pense être au rendez-vous de juillet malgré la complexité technique du dispositif, craint cependant d'être débordée par les demandes d'explications des allocataires et de ne pas être en mesure de les traiter dans des délais raisonnables. L'article 74 de ce PLF rétablit partiellement l'APL accession, dans certaines conditions, mais en outre-mer uniquement. Nous nous en réjouissons, mais, monsieur le ministre, c'est sur l'ensemble du territoire et de manière pérenne qu'il faudrait la rétablir. Je vous proposerai symboliquement un amendement en ce sens. Quant au programme 135, « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », son contenu ne change pas de manière considérable, si ce n'est que 2019 restera l'année de

Un point, maintenant, sur les conséquences de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité, dont le rendement pour l'État, du fait de la baisse des APL, est plus important que prévu : environ 870 millions d'euros en année pleine, contre 800 millions initialement prévus, ce qui signifie que, pour les bailleurs sociaux, le coût est lui aussi plus élevé.

Combien cette hausse de TVA aura-t-elle rapporté en 2018 ? En tout état de cause, nous souhaitons une révision des paramètres pour 2019, afin de rester dans l'objectif prévu de 1,5 milliard d'euros- 800 millions d'euros de réduction d'APL pour financer la RLS, côté dépenses,

de l'action n° 04 en faveur de la Corse, le retard constaté a conduit à prolonger l'action, et des crédits sont ouverts, pour 2019, au même niveau que pour

Le programme 112 s'intitule « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement des territoires ». Or, aujourd'hui, il ne remplit plus cette mission. Son rôle est devenu trop flou, ses missions parfois fluctuantes, et trop d'incertitudes pèsent sur son avenir. Je voudrais illustrer mon propos par quelques exemples. Premièrement, on constate la diminution constante des crédits affectés à ce programme : à l'exception de la seule année 2017, les crédits du programme 112 sont en diminution constante depuis dix ans ; pour la seule période 2011-2019, ils ont chuté de 40 %. Deuxièmement, on note l'affaiblissement des outils de contractualisation. Il y a seulement deux ans, le programme 112 rassemblait les quatre outils financiers de contractualisation avec les territoires : les CPER, ou contrats les contrats État-métropole, les contrats de ville et les contrats de ruralité. Aujourd'hui, deux d'entre eux seulement subsistent dans ce programme, les CPER et les contrats de ville, alors que la politique des territoires mérite une approche globale et cohérente.

Ils l'ont été en 2017, avec des crédits dédiés à hauteur de 216 millions d'euros inscrits au titre du programme 112- c'était cohérent. En 2018, leur financement a été transféré au programme 119, avec seulement 45 millions d'euros de crédits fléchés- ce n'était déjà plus cohérent. En 2019, aucun crédit n'est dédié aux contrats de ruralité, dans aucun programme ! Comment rendre lisible une politique d'aménagement du territoire et comment bâtir des stratégies de développement local dans de telles conditions ? Comment expliquer cette régression aux élus ruraux ? C'est tout simplement impossible ! Enfin, on observe la quasi-disparition de la prime à l'aménagement du territoire. Cette aide directe aux PME vise à soutenir l'emploi dans les territoires les plus fragiles.

ces quelques exemples suffisent à mettre en évidence l'urgence qu'il y a à repenser une nouvelle politique d'aménagement du territoire et à définir la place que l'on veut donner au programme 112 au sein de cette nouvelle politique de l'État. politique de l'État. La récente création de l'agence nationale de la cohésion des territoires nous en donne, je le crois, une occasion unique. J'ai défendu la création de cette agence. Elle a ouvert de nouvelles perspectives, mais les élus attendent désormais qu'elle soit rapidement rendue opérationnelle et qu'elle apporte des réponses efficaces aux besoins de la ruralité. Permettez-moi de soulever, en la matière, quelques questions. Dans quel délai

Cette solution nécessiterait de reconsidérer les crédits alloués à ce programme. Le contrat unique de cohésion territoriale que vous envisagez est-il destiné à se substituer à tous les contrats existants : les CPER, les contrats de ville, les contrats État-métropole, les contrats de ruralité ? Si oui, dans quel délai ?

que les besoins en termes de personnel ne sont pas encore définis ? Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez donner. S'agissant du vote, ces deux programmes représentent seulement 1,7

avis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits des programmes 177, 109 et 135 relatifs au logement diminuent pour la deuxième année consécutive, pour atteindre 15 milliards d'euros. La baisse de 8 % des crédits du programme 109 résulte, d'une part, des mesures d'économies adoptées l'an dernier- suppression de l'APL accession, gel des barèmes et des loyers, soit 222 millions

et qui nécessitera de bien informer les allocataires. Les paramètres de la RLS ont été établis en 2018 pour permettre une économie de 800 millions d'euros Ces paramètres n'étant pas modifiés, la RLS permettra 873 millions d'économies en 2019, soit 73 millions de plus En outre, le rendement de TVA sur les constructions de logements sociaux devrait s'avérer plus favorable et atteindre 850 millions au lieu de 700 millions. Ces économies supplémentaires ne sont pas anodines. Le coût de la RLS pour les bailleurs sociaux est plus important que le montant des économies pour l'État 830 millions en 2018 et 916 millions en 2019. Sans tenir compte des mesures de soutien, la RLS devrait conduire pour 2018 à une perte d'autofinancement nette de 21 et à une baisse de 5 % de la construction de logements sociaux, baisse qui pourrait atteindre 38 % dans vingt ans selon la Caisse des dépôts et consignations. En ne modifiant pas les paramètres de la RLS, le Gouvernement ne respecte pas ses engagements en termes de trajectoire financière. C'est pourquoi la commission des affaires économiques a proposé de rejeter les crédits du programme 109.

S'agissant du programme 135, sans surprise, l'État se désengage définitivement des aides à la pierre, laissant les bailleurs sociaux financer la quasi-totalité des ressources du FNAP. un mot de l'ANAH. Je salue l'augmentation de ses ressources, mais je regrette le manque d'ambition et les contradictions du Gouvernement, qui a préféré plafonner les ressources de l'Agence plutôt que d'utiliser les ressources supplémentaires issues des quotas carbone pour accélérer la rénovation énergétique des logements. logements. Les crédits du programme 177 augmentent à périmètre constant. Malgré un effort de sincérité budgétaire et une rationalisation des coûts, il n'est pas sûr que

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits du programme 147, « Politique de la ville », sont en augmentation de 57 % en autorisations d'engagement et de 19,7 % en crédits de paiement. Nous sommes nombreux à craindre que ces crédits ne soient pas entièrement consommés, les dispositifs financés- je pense à des postes d'ATSEM, à des postes FONJEP ou à des postes d'adultes-relais -supposant bien souvent des cofinancements de la part des associations ou des collectivités territoriales. Or, dans un contexte budgétaire contraint, il n'est pas certain que ces dernières puissent apporter leurs concours financiers ou du moins des financements à la hauteur de l'effort consenti par l'État. Comment peut-on en effet leur demander de consacrer plus de 100 millions d'euros à de nouveaux postes alors que les subventions de l'État sont en baisse ? Quant aux crédits de droit commun, ils peinent à se déployer. La révision des contrats de ville sera l'occasion de vérifier si l'État respecte les engagements qu'il a pris dans le cadre du pacte de Dijon. Après une année d'arrêt, le nouveau programme national de renouvellement urbain semble enfin démarrer. Que de temps perdu ! Si l'on peut se féliciter de la multiplication des signatures de protocoles, je crains néanmoins que les « grues » ne soient pas présentes dans les quartiers avant 2020.

Enfin, il faudra être attentif aux effets des récents choix gouvernementaux en matière d'habitat, tels que la réduction du loyer de solidarité et l'intégration de l'EPARECA au sein de la future agence nationale de la cohésion des territoires.

intégrées. Le programme 147 consacre 101 millions d'euros au développement économique et à l'emploi. La réforme des contrats aidés et l'expérimentation des emplois francs mises en oeuvre l'an dernier n'ont pas produit les effets escomptés et le chômage des jeunes est reparti à la hausse. En matière d'emplois francs, les résultats sont très loin des objectifs fixés. Au 16 septembre septembre 2018, 1 980 demandes d'emplois francs ont été transmises à Pôle emploi et 1 528 ont été acceptées. Je regrette qu'on attende la fin de l'expérimentation avant de corriger le dispositif étant donné que 25 000 demandes sont prévues pour 2019. Le nombre de contrats aidés dans sa nouvelle version est en très forte diminution en raison de l'aspect plus contraignant du nouveau dispositif et d'une moindre prise en charge. Certains préfets n'ont d'ailleurs pas jugé opportun de moduler l'aide pour soutenir le déploiement des contrats dans les quartiers, ce que je regrette. le dispositif manque sa cible en laissant de côté les personnes « employables rapidement » tout en n'étant pas adapté aux personnes les plus éloignées de l'emploi, qui ont besoin d'un temps d'accompagnement plus long. La commission des affaires économiques s'en remet donc à la sagesse du Sénat pour le vote des crédits du programme 147 et a émis un avis favorable sur l'adoption de l'article 74.

la commission des affaires sociales a examiné les crédits du programme 177 de la mission « Cohésion des territoires », qui financent l'hébergement des personnes en détresse et l'accompagnement des plus précaires vers l'accès au logement. Les demandes d'hébergement ont considérablement augmenté ces dernières années, sollicitant fortement les structures financées par le programme- le nombre de places en hébergement d'urgence a progressé de 180 % depuis 2010. En parallèle, les moyens alloués au programme ont augmenté de 562 millions d'euros en cinq ans, soit une hausse de 42 %, ce qui est à souligner dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques. Malgré cette progression, le programme souffre d'une sous-budgétisation chronique, et le recours aux décrets d'avance ou à l'ouverture de crédits supplémentaires en loi de finances rectificative a été systématique ces dernières années. Même si un important effort de sincérité budgétaire a été engagé depuis l'an dernier, l'exécution du programme en 2018 devrait dépasser les 2 milliards d'euros et excéder de 8 l'enveloppe de crédits ouverte en loi de finances initiale. Soulignons cependant que l'écart entre les crédits votés et les crédits exécutés se réduit par rapport aux années précédentes. les crédits demandés s'élèvent à 1,88 milliard d'euros en crédits de paiement. Supérieurs à ceux consommés en 2017, ils restent inférieurs à la prévision d'exécution pour 2018, au risque d'une nouvelle sous-budgétisation en 2019. Le budget du programme s'inscrit dans le cadre du plan Logement d'abord et de la stratégie de lutte contre la pauvreté annoncée en septembre dernier, dont les orientations sont approuvées par la commission des affaires sociales. Elles visent à développer les modes de logement adapté et les structures d'hébergement des familles, ainsi qu'à renforcer les dispositifs de veille sociale. Les crédits sont certes en augmentation pour mettre en oeuvre ces orientations, mais ils n'apparaissent pas suffisants pour atteindre les objectifs fixés. Concernant le logement adapté, l'objectif de doubler le nombre de places en cinq ans dans l'intermédiation locative et en pensions de familles sera difficile à atteindre avec seulement 8,4 millions d'euros supplémentaires alloués à ces deux dispositifs en 2019. Ce sont surtout les moyens dédiés à l'accompagnement social qui ne semblent pas suffisants. Sur ce point, les mesures annoncées par le Gouvernement vont dans le bon sens : renforcement des maraudes, accompagnement pour la sortie de l'hébergement à l'hôtel, création de référents de parcours pour un meilleur suivi de la personne. Sauf que les financements de ces dispositifs ne sont pas bien identifiés, voire pas encore prévus ! Le plan de limitation des nuitées d'hôtel a certes permis de contenir leur progression, mais ce mode d'hébergement continue de croître. Le plus préoccupant est que l'hôtel perd progressivement sa vocation d'hébergement temporaire pour accueillir des personnes pendant plusieurs années. En outre, certaines grandes agglomérations voient dorénavant leur capacité hôtelière saturée. Un accompagnement social renforcé doit permettre d'assurer une meilleure rotation des publics accueillis afin de répondre aux situations de détresse. À cet égard, le plan d'économies de 57 millions d'euros imposé aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale sur trois ans fragilise l'accompagnement social qu'apportent ces structures. Si l'objectif du plan Logement d'abord vise à trouver une solution de logement sans passer systématiquement par des structures temporaires, il ne peut être atteint à court terme en affaiblissant les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Malgré les insuffisances dont je viens de vous faire part, la commission des affaires sociales a tenu à saluer l'effort de sincérité budgétaire et les orientations prises en faveur de l'hébergement et de l'accès au logement. C'est pourquoi elle a donné un avis favorable sur l'adoption du programme 177. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a rendu un avis défavorable l'adoption des crédits des programmes 162 et 112 de la mission « Cohésion des territoires » et des crédits du compte d'affectation spéciale consacré au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale. Plusieurs raisons justifient ce choix. En premier lieu, la commission considère que la trajectoire de ces crédits n'est pas compatible, en l'état, avec le projet de création de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, vous nous préciserez sans doute que les conséquences budgétaires de la création de cette agence, qui a été initiée par le vote de deux propositions de loi, l'une ordinaire, l'autre organique, au Sénat le 8 novembre dernier, seront tirées dans le projet de loi de finances pour 2020, mais je souhaitais rappeler ce point. deuxième lieu, s'agissant du programme 112, la commission a déploré l'érosion continue de la prime d'aménagement du territoire. Le montant de ce dispositif est certes modeste, mais il joue un rôle d'entraînement important dans les territoires et permet de renforcer leur l'attractivité. Aussi, je salue l'initiative du rapporteur spécial Bernard Delcros, qui proposera tout à l'heure un amendement à l'article 39 visant à augmenter de 5 millions d'euros les autorisations d'engagement profit de la PAT, afin de stabiliser les moyens engagés à hauteur de 15 millions d'euros, comme en 2018. Au-delà de ces observations, j'ai deux interrogations. La première concerne le plan chlordécone, porté par l'action n° 08 du programme 162, « Interventions territoriales de l'État ». Le Président de la République était aux Antilles en septembre dernier, et il a eu des mots que je qualifierais de courageux et qui l'honorent, mais qui l'obligent également après avoir expliqué que l'État prendrait « sa part de responsabilité » dans ce scandale environnemental et sanitaire, le Président de la République a annoncé une augmentation des moyens consacrés à ce plan à hauteur de 3 millions d'euros sur deux ans.

Le Sénat propose depuis plusieurs années une évolution de son dimensionnement et de sa gestion pour l'adapter aux enjeux de la transition énergétique, car les communes rurales ont besoin de soutien en matière environnementale. Je souhaiterais que le ministère de la transition écologique précise ses intentions sur ce sujet. Mes chers sur ce sujet. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, en ces temps où l'on parle beaucoup trop de divisions dans notre société, je tiens à rappeler combien je suis heureux d'être parmi vous et d'intervenir dans ce débat sur la cohésion des territoires, avec des élus issus de toute la diversité des territoires et des structures administratives de notre pays.

Il ne s'agit en rien d'opposer des France entre elles, mais il faut permettre à chacune de suivre sa propre trajectoire de développement, sous le socle de valeurs et de lois communes, dans le respect des identités et des possibilités de chacun, au sein de la République une et indivisible. Dans ce budget, le groupe du RDSE a souhaité donner plus de visibilité et d'efficacité à des axes qui nous tiennent à coeur : la réhabilitation des centres-villes, la création de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Nous avons ainsi déposé plusieurs amendements visant à renforcer le plan « Action coeur de ville » et à l'adapter au mieux à la réalité des situations. Nous proposons de favoriser l'investissement dans les centres-villes, plus particulièrement pour les logements de taille moyenne, d'augmenter des dispositifs de réduction fiscale afin de répondre au montant réel du coût des travaux de réhabilitation de l'ancien et d'inclure la transformation de locaux en logements dans ces mêmes centres-villes. Concernant la création prochaine de l'agence nationale de la cohésion des territoires, je suppose que vous comprendrez, monsieur le ministre, que nous sommes inquiets sur le montant des crédits alloués au programme 112. Celui-ci, en diminution continue, n'est pas compatible avec l'ambition de la création de l'agence que le Gouvernement a soutenue et appuyée. Nous rappelons, de plus, que l'agence doit pouvoir, dès sa création, être aussi pleinement efficiente pour les territoires ruraux et périurbains, alors que l'intégration des programmes 112 et 147 fait craindre le contraire. Nous insistons à ce titre sur le risque de dissolution de crédits spécifiques à la ruralité dans le contrat de cohésion territoriale. Nous pensons, enfin, qu'il n'est pas opportun de diminuer des postes du CGET au moment même de la création de l'agence nationale. Cette agence n'est pas qu'un outil facilitant la gestion administrative, mais est une agence de service public, avec des moyens humains dédiés. Monsieur le ministre, la dématérialisation ne peut se faire partout, uniformément, de la même manière. Nombre de nos concitoyens et nombre d'élus sont confrontés à un changement d'échelle de responsabilité, mais aussi à un changement trop radical de culture administrative qui altère la perception du service public, il faut le dire. Nous devons veiller à ce que le rythme de réforme soit adapté et ne laisse personne sur le bord du chemin. Je terminerai mon propos par une remarque qui dépasse les frontières de ces budgets. La cohésion des territoires, c'est la liberté pour tout citoyen français de s'installer où il veut, quand il veut et d'y trouver les mêmes droits, les mêmes services qui fondent l'égalité républicaine. l'égalité républicaine. Ce budget permet d'adopter des mesures qui seront visibles à moyen ou à court terme. Cependant, sans couverture mobile partout, sans couverture numérique minimale, ces investissements seront un tonneau des Danaïdes que la solidarité nationale n'aura pas fini de remplir Mes chers collègues, le mobile, le numérique partout, c'est la garantie que les mesures que nous votons pourront vraiment changer la vie quotidienne de nos territoires. Vous me permettrez d'être concret : un artisan en zone hyper rurale sans haut débit ne peut accéder aux appels d'offres pourtant baissés à 25 000 euros. Où est l'égalité républicaine ? Quand un collège en bas débit ne peut organiser décemment des examens pour ses élèves et charge un conseil départemental de trouver un bus scolaire pour amener ces enfants dans un collège disposant du débit suffisant, où est l'égalité républicaine et où est l'autonomie des collectivités territoriales ? Quand une mairie charge un employé d'aller chercher en catastrophe dans une sous-préfecture la liste d'émargement nécessaire à des élections faute de haut débit, où est l'égalité républicaine, où est l'autonomie des collectivités territoriales ? Monsieur le ministre, l'équipement mobile et numérique peut être accéléré dès maintenant. Nous devons disposer des arrêtés permettant l'intervention des opérateurs dans les plus brefs délais. Nous devons et pouvons utiliser dès dès maintenant les pylônes TDF pour les rendre opérationnels. La cohésion des territoires peut aussi s'écrire dans le court terme. Les zones oubliées, blanches ou grises, constituent des leviers de croissance et de développement sous-estimés. Bravo ! La parole

Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens ! Oui, la France est riche de sa diversité Chirac exprimait cette nécessité d'assurer la cohésion de nos territoires, de réduire les disparités sociales et territoriales tout en préservant les spécificités et les richesses de la France. C'était le La mission « Cohésion des territoires » est importante, du fait de la transversalité des sujets évoqués et des actions menées dans les six programmes concernés. Elle doit contribuer à mettre en en place un aménagement équilibré, garant de la cohésion, de la performance et de la solidarité territoriale. Nous devons donc investir dans un projet de cohésion de nos territoires fort, avec des outils performants au service de nos collectivités. En ce sens, nous pouvons saluer la hausse de près de 20 % du budget consacré à la politique de la ville du programme 147, politique importante pour réduire les inégalités entre les quartiers populaires et les autres territoires. Ces crédits supplémentaires devront être fléchés de façon pertinente, en lien avec les priorités des collectivités locales. Sur ce programme, le retard du démarrage du nouveau programme national de renouvellement urbain est regrettable. Nous espérons que sa mise en oeuvre avec toutes les parties concernées sera accélérée et que le doublement de son budget au profit de l'ANRU se traduira par des réalisations concrètes dans nos territoires. Nous saluons la rationalisation du calcul des aides personnalisées au logement du programme 109, qui se fera sur la base de la situation actuelle des revenus déclarés, et non plus à n-2. Cela semble plus juste et plus simple. Dans le programme 112, « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », on ne peut que regretter l'absence de financement dédié aux contrats de ruralité et leur retrait du programme. Nous serons extrêmement vigilants à la prise en compte des enjeux ruraux dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de cohésion territoriale porté par la future agence nationale de la cohésion des territoires. Il faut absolument éviter une dissolution des moyens mis en place pour nos territoires ruraux. Nous devons veiller à ce que la contractualisation avec les territoires conduise bien à soutenir les projets prioritaires des collectivités territoriales, que ce soit au travers des contrats de plan État-régions 2015-2020, des dotations de soutien à l'investissement public local ou des dotations d'équipement des territoires ruraux. Alors que l'accès au numérique et les maisons de services au public sont deux dossiers prioritaires pour réduire les fractures territoriales, notamment dans nos communes rurales, le programme « Action coeur de ville » doit permettre de redynamiser les centres-villes et de renforcer leur attractivité. Par ailleurs, nous sommes inquiets de la baisse de la prime d'aménagement du territoire. Nous avons déposé un amendement visant à revenir à la situation de 2018, avec une stabilisation de la dotation à 14,5 millions d'euros en autorisations d'engagement. Il s'agit de réfléchir à une refonte en profondeur du dispositif. Il convient, plus largement, de s'interroger sur la compatibilité de l'amenuisement des crédits du programme 112 avec la création prochaine de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Sur le programme 135, « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », le budget priorise la rénovation des logements, avec un budget de 110 millions d'euros pour l'Agence nationale de l'habitat et une hausse de 40 millions d'euros de la taxe sur les logements vacants qui lui est affectée. Il nous semble important de soutenir cette agence pour maintenir la qualité et l'ambition du programme « Habiter mieux », reconnues par la Cour des comptes, en lui fournissant les moyens nécessaires à son action. Nous saluons la reconduction pour quatre ans des dispositifs Pinel et du prêt à taux zéro afin de donner une meilleure visibilité aux acteurs concernés. Par ailleurs, nous regrettons que la contribution de l'État au budget du Fonds national des aides à la pierre soit supprimée. C'est un programme important pour la construction de logements sociaux pour lequel les besoins des collectivités locales doivent être mieux pris en compte par les bailleurs sociaux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants-République et Territoires s'abstiendra donc sur les crédits de cette mission.

Présenter un budget en diminution pour 2019- s'agissant pour l'essentiel d'une moindre dépense d'aides au logement -n'est pas un manque d'ambition ou un désengagement des pouvoirs publics. Au contraire, c'est le choix de l'efficacité dans un secteur qui est tout à la fois une préoccupation majeure de nos concitoyens, un secteur clé de notre économie et, reconnaissons-le, un synonyme d'échec. Un échec coûteux, financièrement, puisque 40 milliards d'euros sont engagés chaque année sur le logement. un échec sur le plan social, puisque la Fondation Abbé-Pierre estime à près de 4 millions le nombre de nos concitoyens en situation de grande précarité en matière de logement. En un mot, en matière de politique du logement, il n'y a pas toujours eu de corrélation nette entre crédits budgétaires et crédibilité politique. En France, on pratique souvent la critique des réformes en oubliant parfois le diagnostic de départ, comme si auparavant loi de finances pour 2019 prévoit de mettre en oeuvre la réforme du calcul des allocations logement. C'est un sujet qui a été maintes fois évoqué, mais, monsieur le ministre, vous transformez l'essai. Le calcul contemporain des ressources des APL, c'est tout à la fois une mesure de justice et d'économie, puisque 900 millions d'euros sont attendus de cette réforme. Dès l'an prochain, l'éligibilité d'un demandeur aux APL sera calculée non plus en fonction de ses ressources n-2, mais sur la base des douze derniers mois, grâce à une base de données alimentée par le prélèvement à la source. J'ai entendu les réserves émises par le rapporteur spécial Philippe Dallier quant à la faisabilité de cette réforme et sur le montant des économies dégagées par sa mise en oeuvre. Cette réforme demandera de l'agilité, car les APL seront recalculées chaque trimestre, et de la fluidité puisque les échanges de données entre la CNAF et les services de la DGFiP seront essentiels pour déterminer les ressources des ayants droit. Elle demandera aussi de la publicité à travers une communication claire pour les bénéficiaires comme pour les bailleurs. Dans un contexte de rareté de l'argent public, il me semble essentiel d'allouer les APL à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le nouveau mode de calcul permettra également de réduire le niveau de non-recours, car il est choquant que des personnes ne fassent pas valoir leurs droits.

L'émancipation des jeunes passe par le logement. Leur désir d'autonomie est parfois contrarié par le prix élevé du logement. Une étude de 2016 estime, par exemple, que sept jeunes de dix-huit à trente ans sur dix déclarent avoir déjà éprouvé une difficulté à se loger. Le bail mobilité est un nouveau type de contrat, d'une durée de un à dix mois. Il concerne les logements meublés et s'adresse en priorité aux étudiants, aux personnes en formation, en mutation ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle. Il sera sans dépôt de garantie, mais il sera sécurisé par la garantie gratuite Celle-ci est un dispositif simple et dématérialisé, qui couvre jusqu'à trois ans d'impayés. Le public cible est large : jeunes de moins de trente ans, salariés de plus de trente ans sans CDI confirmé et les ménages en intermédiation locative. Dans le parc social, 80 000 logements seront construits à destination des jeunes d'ici à 2022, 60 000 logements étudiants et 20 000 logements pour les jeunes actifs. J'appelle de mes voeux des actions de communication offensives pour bien faire connaître ces nouveaux dispositifs. L'élu parisien que je suis ne peut qu'être sensible à l'encadrement des locations touristiques. En effet, les contrôles et les sanctions, en matière de location courte durée, seront renforcés à l'encontre des loueurs et des plateformes qui ne respectent pas la loi. La location de la résidence principale est limitée à 120 nuitées par an, mais celle des résidences secondaires dépend des territoires. La question reste devant nous pour la capitale, toute la capitale, pas uniquement les arrondissements du centre. Il est important de prévoir des garde-fous, tout en gardant à l'esprit que c'est un moyen pour des ménages de « mettre du beurre dans les épinards En tout cas, les sanctions pourront aller jusqu'à 10 000 euros par logement pour les propriétaires et à 50 000 euros pour les plateformes. Il est important d'avoir accru ces sanctions, car la mesure était attendue dans les villes. La loi ÉLAN permet également d'apporter des réponses concrètes à des déséquilibres territoriaux. C'est, par exemple, la transformation des bureaux en logements. En Île-de-France, les professionnels estiment que près de 700 000 mètres carrés de bureaux sont obsolètes et durablement vacants. Le bénéfice est clair : c'est un gisement potentiel de 10 000 à 20 000 logements pour la région. C'est aussi surtout le plan « Action coeur de ville », qui prévoit de redonner de l'attractivité à 222 villes moyennes en matière d'habitat, de commerce, de transports. Cette préoccupation se retrouve d'ailleurs dans l'article 74 instaurant une réduction d'impôt pour l'investissement dans les logements locatifs intermédiaires réhabilités en centres-villes. Cela permet de sortir des guerres picrocholines du zonage de la politique du logement, qui, objectivement, manque de lisibilité et d'efficacité. Cela permet également de mettre de la cohérence entre le dispositif « Action coeur de ville » et ce dispositif. L'engagement du Gouvernement en faveur de l'hébergement est total. Monsieur le ministre, je tiens à vous redire publiquement le soutien du groupe La République En Marche sur le plan Hiver déployé depuis le 1 novembre dernier pour mettre à l'abri les personnes dans cette période critique. 6 millions d'euros sont fléchés pour le soutien des maraudes, essentielles pour identifier les situations de fragilité. Par ailleurs, 105 000 personnes sont hébergées chaque soir en Île-de-France. L'objectif de l'État est de trouver 7 000 places cette année en Île-de-France, dont 3 700 à Paris. Enfin, je ne peux conclure mon propos sans dire un mot de l'habitat indigne et dégradé, qui a été mis en évidence par le drame de Marseille. C'est le sens de l'initiative « copropriétés », qui mobilisera 3 milliards d'euros qui sont les plus dégradées. C'est surtout l'accélération de la rénovation urbaine : le budget de l'ANRU est doublé de 5 milliards à 10 milliards d'euros, le taux de subvention pour la démolition des copropriétés très dégradées passe de 50 % à 80 % et l'accompagnement des élus est renforcé pour simplifier la conduite des projets. J'ai entendu aujourd'hui beaucoup de critiques dans les interventions. Parfois, la force des propositions n'est pas en rapport avec vigueur de ces critiques. Je pense, notamment, aux nombreux amendements budgétaires qui tendent

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de cette mission sont très vastes, puisqu'ils recouvrent les crédits de deux anciens programmes : la politique des territoires et le logement. Je ne pourrai donc pas, dans le temps qui m'est imparti, être exhaustif ; il y aurait pourtant beaucoup à dire. Quelques mots tout de même sur le lien entre les élus et l'État, marqué par la défiance et le mépris. En témoigne l'absence du Président de la République au Congrès des maires qui s'est tenu la semaine dernière. En témoigne également la poursuite des politiques marquées du sceau de l'austérité, qui renforcent les inégalités territoriales. L'État organise aujourd'hui sa propre faillite en se privant de compétences avec la baisse généralisée des moyens, humains et financiers, au sein de ses services, agences et opérateurs. Conjuguée à la baisse continue des dotations aux collectivités, les conséquences concrètes en matière de service public seront dramatiques. Je pense ici particulièrement aux habitants des territoires ruraux, des outre-mer, mais également des banlieues, qui attendaient beaucoup du plan Borloo, jeté aux oubliettes dès sa parution. sa parution. Les politiques publiques ne font office que de rustines inefficaces, alors que les maux sont très lourds : concentration du chômage, des difficultés scolaires et de logement, difficulté de mobilité, d'accès aux loisirs et à la culture, autant de chantiers que vous ne voulez pas affronter, préférant faire des cadeaux à la finance. C'est un choix politique que nous ne partageons pas, considérant que concurrence et libéralisme ne font pas bon ménage avec aménagement du territoire et maintien des services publics. En matière de droit au logement, l'année qui vient de s'écouler a été particulièrement difficile, marquée par l'accroissement des expulsions locatives, par des morts dans la rue faute de place dans les structures, par la baisse des APL, par les scandales de l'insalubrité, qui ont conduit à l'effondrement d'immeubles, comme récemment à Marseille, et, enfin, par l'adoption de la loi ÉLAN, un pas supplémentaire vers la financiarisation et la privatisation du logement social, confirmant ainsi le désengagement de l'État. La Seine-Saint-Denis est particulièrement touchée par l'insalubrité, vous le savez, monsieur le ministre. À Aubervilliers, où vous avez effectué une visite avec sa maire,

qui, pour la première fois, ne s'engage plus dans les aides à la pierre : zéro euro pour la construction ! Déjà, depuis l'an dernier, il n'apportait plus son aide aux maires bâtisseurs. Une décision symbolique, alors même que la loi SRU a été largement remise en cause par la loi ÉLAN. À l'inverse, les dispositifs de soutien à l'investissement locatif entraînent une dépense fiscale toujours plus importante, de l'ordre de 1,3 milliard d'euros sur les 13 milliards de dépense fiscale générale liée à ce programme. Nous considérons, pour notre part, qu'il convient, au regard de l'ampleur des sommes en jeu, d'opérer une véritable analyse sur l'efficacité de cette dépense, laquelle serait bien plus utile pour soutenir directement la production sociale et l'effort de rénovation du parc public comme du parc privé. Disons-le, mes chers collègues, l'insalubrité et les marchands de sommeil sont le revers d'un marché saturé par la demande, où le logement est à la fois rare et cher. Avec la loi ÉLAN, les conséquences sur la construction seront dramatiques. Ainsi, selon une étude de la Caisse des dépôts et consignations, les baisses de crédits et les changements de modèle vont conduire à pénaliser la construction, alors que l'on recense plus de 2 millions de demandeurs de logement. À court terme, le secteur se maintiendrait grâce à sa solidité et à la vente des logements sociaux, mais, à long terme, ce serait la catastrophe. Dès 2020, la production passerait sous la barre des 100 000 logements construits, puis se situerait à une moyenne de 63 000 entre 2027 et 2055. Seulement 63 000, alors que ce sont 200 000 logements sociaux qu'il faudrait construire par an pour répondre à la demande sociale d'un renoncement de l'État, lequel doit pourtant garantir le droit constitutionnel d'accès au logement pour toutes et tous dans des conditions abordables. La soutenabilité même du système nous inquiète, alors que nous savons tous que le secteur HLM sera incapable de faire face à la deuxième étape de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité, prévue pour 2020. Vous demandez un effort impossible, qui va conduire à stopper la construction et à brader aux investisseurs privés le parc existant.

qui a transféré la charge de ces aides aux bailleurs pour 873 millions d'euros, par la suppression des APL accession pour 70 millions d'euros et le gel des prestations pour 126 millions d'euros. Et pourtant,

soit une économie cumulée de plus de 2 milliards d'euros sur le dos des plus fragiles, pour aider les multipropriétaires à acquérir de nouveaux biens les dispositifs d'aide à l'investissement locatif. Comme toujours avec ce gouvernement, c'est sur le dos des plus fragiles, de ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, que cette économie va se faire ! Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas ces crédits, très faibles, qui témoignent d'une volonté de casser un modèle social- unique en Europe, voire dans le monde -pourtant performant, de s'affranchir de toute idée de solidarité nationale, alors que même la Commission européenne appelle les États membres à réinvestir dans ce secteur. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

en matière de stratégie de logement, qui se situe dans la continuité assez logique de notre dernier débat budgétaire. Les crédits de la mission « Cohésion des territoires » sont de nouveau en baisse, une diminution liée à la poursuite des mesures de réduction des aides personnalisées au logement et de refonte de leur mode de calcul. APL comptent pour 82 % de ce budget. En effet, les crédits du programme 109, « Aide à l'accès au logement », sont en nette diminution entre 2018 et 2019, passant de 14,26 milliards à 13,11 milliards d'euros, soit une baisse de 8 %. Outre que ce budget nous laisse un sentiment de déjà-vu, il nous confirme que les APL restent une variable d'ajustement budgétaire, avec cette baisse de 1,2 milliard d'euros qui est la conséquence de plusieurs décisions. la non-indexation de l'APL sur l'inflation, pour une économie de 102 millions d'euros, remplacée par une revalorisation de 0,3 %, qui risque de créer un effet ciseaux regrettable, couplé avec le prélèvement à la source. la réforme du mode de calcul de l'APL, pour 910 millions d'euros d'économies. À ce titre, permettez-moi de m'interroger doublement. Je ne comprends pas que l'on ait préalablement fait le choix de la baisse des APL avant d'en modifier le mode de calcul. Par ailleurs, concernant le calcul sur la base des revenus actuels de l'allocataire- la contemporanéisation -, les difficultés qui s'annoncent vous ont fait finalement prévoir une entrée en vigueur au premier semestre de 2019,

Enfin, la mise en oeuvre de la RLS, concomitamment avec la baisse des APL, tend à produire les effets que nous craignions et sur lesquels nous vous avions longuement alerté l'an passé. Vous avez demandé un effort important aux bailleurs sociaux- 800 millions d'euros en 2018 -, avec l'idée d'une trajectoire identique en 2019. Entrée en vigueur au 1 février 2018, cette économie a donc été réalisée en onze mois. Si, aujourd'hui, les paramètres ne sont pas modifiés, la RLS représentera pour l'année 2019 un coût de 873 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, soit 73 millions de plus que ce qui était prévu dans la trajectoire initiale. Aussi, les membres du groupe Union Centriste,

comptez-vous éviter ces effets de bords et faire en sorte que les bailleurs sociaux ne soient pas sollicités au-delà de ce qui était nécessaire ? Le rendement de la TVA sur les constructions de logements sociaux s'annonce par ailleurs supérieur à ce qui était envisagé et pourrait atteindre 850 millions d'euros en 2019. Sur ce sujet, nous suivrons

Il ne me semble pas que nous puissions faire l'économie d'un mot sur la situation des bailleurs, qui, avec la mise en place de la réforme, couplée à la restructuration du secteur prévue dans la loi ÉLAN, sont exsangues. Une perte d'autofinancement net de 21 % est constatée sur l'année 2018. Le nombre d'organismes en situation de fragilité passerait

En 2018, sur un objectif de production de 2 000 logements sociaux dans la métropole de Lille, on constate une réduction des constructions de 600 logements, alors même que le fait d'être dans une métropole devrait faciliter le dispositif. Quand bien même les bailleurs sociaux ont les moyens de trouver des financements, ils ont besoin d'avoir des fonds propres. Le secteur du logement social connaît de grandes difficultés, avec probablement moins de 100 000 logements financés, contre 126 000 en 2016 et 113 000 en 2017. Les chiffres concernant le nombre d'organismes en grande difficulté ou en autofinancement négatif sont de plus en plus inquiétants. En l'état actuel, et avec les mêmes conditions de financement, les ESH ne sont pas exemptées de ces problèmes, puisque leur taux d'autofinancement courant devrait être pratiquement divisé par trois en trois ans et pourrait devenir négatif à partir de 2025. Ce sont 28 nouvelles ESH qui passeraient dans le rouge dès 2018.

et nous sommes nombreux sur ces travées à vous avoir alerté sur ce point, que l'effet inverse ne se produise. De mois en mois, la construction de logement diminue. Les mises en chantier de logements neufs ont ainsi reculé de 7,9 % au troisième trimestre. Il est à craindre que moins de 400 000 logements soient construits en 2019, et nous constaterons sans doute une perte de 40 000 logements en raison des restrictions du prêt à taux zéro, du dispositif Pinel, de l'APL accession et de la baisse des commandes HLM. La dégradation du secteur du logement impactera fortement nos territoires, avec des écarts

Nous suivrons Philippe Dallier dans son souhait de rétablir l'APL accession, et nous vous proposerons au cours du débat des amendements de rééquilibrage du dispositif Pinel, afin qu'il soit adapté aux réalités des territoires en laissant les acteurs locaux responsables du zonage. Nous devons réfléchir collectivement à des dispositifs pour qu'aucun territoire ne soit laissé en marge. Au-delà de la situation du logement, et s'agissant des autres programmes de la mission, nous observons quelques notes positives, non dénuées malgré tout d'interrogations. Concernant le programme « Hébergement d'urgence », nous nous félicitons de la hausse de 43 millions d'euros des crédits de paiements, mais nous sommes

la mission « Cohésion des territoires » couvre l'ensemble des actions mises en oeuvre en faveur du développement et de l'aménagement du territoire, du renouvellement urbain, de la solidarité entre les territoires, du logement, de l'hébergement et de l'habitat durable. Pour l'ensemble de cette mission, 16,1 milliards d'euros sont inscrits en autorisations d'engagement et 16 milliards d'euros en crédits de paiement. Comme l'année dernière, le budget de la mission « Cohésion des territoires » est en baisse : 5,8 pour les autorisations d'engagement et 6,9 % pour les crédits de paiement. Avec une diminution de plus de 1 milliard d'euros, le budget du ministère est mis une nouvelle fois à contribution, dans le cadre de la réduction des dépenses publiques. Tous les postes sont touchés, à l'exception de la politique de la ville. Dans le budget pour 2018, le programme 147, « Politique de la ville », avait accusé une baisse des crédits de paiement de 16 % en autorisations d'engagement, mais les crédits de paiement étaient demeurés stables. Si le Gouvernement n'a pas souhaité reprendre l'ensemble des propositions de Jean-Louis Borloo, il a cependant, en juillet dernier, annoncé un plan de mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, comprenant des mesures en matière de sécurité, d'éducation, d'emploi, de logement, d'amélioration du cadre de vie et de soutien aux associations. Alors, que prévoit le budget pour 2019 ? Devant l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous l'avez qualifié de « deuxième grand pilier de l'action gouvernementale », de « priorité absolue du Gouvernement Effectivement, la politique de la ville semble être la seule rescapée dans un océan de baisses. Conformément aux engagements pris en juillet dernier, les crédits du programme 147, « Politique de la ville », sont en hausse de 244 millions d'euros, de 57 % en autorisations d'engagement, et de 84,4 millions d'euros, soit une hausse de 19,7 %, en crédits de paiement. Si l'on peut se réjouir de cet engagement accru de l'État dans la politique de réduction des inégalités territoriales, il reste toutefois très ciblé. Les actions territorialisées concentrent plus de 62 % des crédits du programme, soit 419,4 millions d'euros à destination des quartiers prioritaires de la mis en oeuvre dans le cadre des contrats de ville ou de dispositifs spécifiques tels que le programme de réussite éducative, ou encore une partie du financement du dédoublement des classes de CP en REP et REP +. L'effort budgétaire porte sur les actions en matière d'éducation et de lien social. prévoit notamment la création de 1 000 postes supplémentaires d'adultes-relais, le doublement du nombre de postes de coordinateurs associatifs, ou encore le renforcement de l'encadrement en maternelle dans une soixantaine de grands quartiers, avec une aide aux communes pour la création de postes d'ATSEM. la politique de la ville est construite autour de la contractualisation. Dans un contexte de baisse des dotations, les collectivités auront-elles les moyens de s'y investir ? Nous ne le pensons pas. S'y ajoute la création d'une nouvelle dotation de 15 millions d'euros pour certaines associations nationales structurantes afin qu'elles soutiennent et mettent en oeuvre des actions de proximité. Le Gouvernement souhaite ainsi soutenir l'emploi associatif. Mais il ne faut pas se leurrer, cette aide ne compense pas la réduction drastique des emplois aidés. Ce sont 20 000 associations qui ont disparu. Quant à l'expérimentation des emplois francs, si les résultats sont loin des objectifs qui étaient affichés, 237 millions d'euros sont pourtant inscrits en autorisations d'engagement et un peu plus de 70 millions d'euros en crédits de paiement. L'augmentation la plus notable du programme concerne l'action n° 04, Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie, qui porte les crédits consacrés au NPNRU. Le budget pour 2018 avait acté le retour de l'État dans le financement du renouvellement urbain, aux côtés d'Action logement et des bailleurs sociaux. Le Gouvernement s'était engagé à porter le NPNRU de 6 milliards à 10 milliards d'euros sur la durée du programme, avec une part de financement de l'État de 1 milliard d'euros, soit 200 millions d'euros par an au cours du quinquennat. Pourtant, en 2018, seuls 15 millions d'euros étaient inscrits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Dans le budget pour 2019, l'État augmente sa participation, qui atteint 185 millions d'euros en autorisations d'engagement et 25 millions d'euros en crédits de paiement. En proportion de son engagement global, l'État finance cependant moins que les bailleurs sociaux et Action logement. L'article 74 du projet de loi de finances acte la participation des bailleurs sociaux au financement du NPNRU, à hauteur de 154 millions d'euros par an pendant toute la durée du programme, soit jusqu'en 2031. La mise en place du NPNRU a accusé des retards : cinq ans après l'adoption de la loi de programmation, les contrats commencent seulement à être signés ... Mais, finalement, ces retards ont permis à l'ANRU de ne pas mettre à mal sa trésorerie. Le groupe Les Républicains est favorable à cet article 74. S'il faut reconnaître que les dépenses du programme 147 relatif à la politique de la ville concrétisent des engagements présidentiels, ces signaux positifs qui se mesurent en millions d'euros ne sauraient masquer les coups de rabot, qui, eux, se chiffrent en milliards.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Commission européenne vient d'appeler les pays européens à investir massivement dans le logement social, afin de faire face à la pénurie de logements abordables, présente dans de nombreux pays. La production de logements sociaux a en effet plongé partout en Europe depuis une dizaine d'années, excepté en France, où elle est restée supérieure à 100 000 logements par an. Beaucoup de pays européens ont mené des réformes, comme le retrait de l'investissement public ou la vente du parc social, dont on voit aujourd'hui les effets désastreux, et ils font maintenant Monsieur le ministre, vous n'allez pas dans le sens de l'Europe, qui invite donc à prendre en compte la crise du logement et à relancer l'investissement public dans « le logement abordable », dont le logement social, le locatif intermédiaire et l'accession à la propriété.

ce sens, contrairement à l'Allemagne, où Mme Merkel vient de lancer son offensive avec un plan volontariste de 5,7 milliards d'euros sur quatre ans pour construire 1,5 million de logements, renforcer les aides et stimuler l'accession à la propriété, contrairement aussi à Theresa May, qui a lancé un plan de 2,3 milliards d'euros dédiés aux collectivités locales et bailleurs sociaux afin de construire et de réhabiliter le parc britannique de logements sociaux. Dans la continuité du budget précédent, votre objectif demeure, en effet, de faire des économies sur le logement. Rappelons que, jusqu'en 2017, notre pays faisait figure d'exception : alors que la production de logements sociaux s'effondrait en Europe, la France construisait encore plus de 100 000 logements sociaux par an. Malheureusement, tous les voyants sont au rouge, avec une production de logements en baisse, comme le prouvent les chutes de 5 % des autorisations de mise en chantier et de 12 % des dépôts de permis de construire, avec les mises en vente qui se contractent fortement, en baisse de 13 %. La diminution des agréments initiée en 2017, en baisse de 9 %, semble se prolonger de 5 % en 2018. Avec vos réformes, la France est à contre-courant. L'affaiblissement des ressources des organismes d'HLM, leur restructuration à marche forcée ainsi que la vente contrainte de leur patrimoine vont sérieusement déstabiliser le secteur. La suppression de l'APL accession, qui représente 50 millions d'euros, et le recentrage du prêt à taux zéro sur les zones tendues ont eu des effets quasi immédiats sur la construction le nombre de permis de construire pour des maisons individuelles a chuté de 14 % par rapport à la même période de 2017. Là où les ménages modestes pouvaient encore accéder à la propriété, les aides ont été supprimées. On est bien loin d'un « élan » du choc de l'offre Pour 2019, le budget dédié à la cohésion des territoires se contracte de 1 milliard d'euros, dont 900 millions d'euros du fait de l'application en année pleine de la RSL, qui a rapporté 800 millions d'euros cette année et dont le Gouvernement escompte 870 millions d'euros l'année prochaine. S'ajoute à cela la contemporanéité des APL. Mais il faudra les moyens nécessaires aux CAF, qui sont vraiment terrorisées par cette nouvelle procédure. Vous poursuivez aussi votre politique d'économies sur les APL, revalorisées à 0,3 % seulement, d'où 102 millions d'économies pour le budget. Si les organismes d'HLM semblent avoir intégré la baisse de leurs ressources en 2018, leur capacité à absorber la montée en charge de la RLS prévue en 2020, avec un quasi-doublement de la ponction- 1,5 milliard d'euros -, suscite de nombreuses inquiétudes.

par ailleurs, quel sera le devenir de l'aide à l'accession à la propriété, que vous rétablissez temporairement et à budget constant au détriment de l'action Urbanisme ? Et où sont les mesures de prévention des copropriétés dégradées dont parlait Valérie Létard ? Je terminerai en évoquant le budget dédié à l'hébergement d'urgence, en hausse de 12 %, ce que nous saluons. Cependant, la situation des CHRS nous inquiète, car cette hausse est fléchée sur les places d'urgence et les nuitées hôtelières. Elle ne bénéficiera donc pas aux CHRS, qui assurent l'hébergement d'insertion. Nous craignons aussi la fermeture de certains centres et de postes d'intervenants sociaux, ce que nous ne pouvons accepter, même si vous avez fléché 20 millions d'euros supplémentaires en direction des sorties de familles des hôtels. Monsieur le ministre, le logement n'est pas une marchandise comme une autre. C'est un toit, c'est un refuge, c'est aussi notre intimité ... Financiariser le logement, c'est accentuer la précarité de milliers de nos concitoyens qui, pour certains, n'arrivent plus à faire face. La vente massive de logements ne saurait compenser la baisse de ressources des bailleurs sociaux. Les questions essentielles aujourd'hui concernent la capacité du secteur du logement social à faire face à l'ensemble des réformes que vous avez décidées, et notamment au « mur » de 2020, et les difficultés toujours croissantes des Français à accéder à un logement « abordable » qui réponde à leurs besoins. Le groupe socialiste votera

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour faire quelques remarques sur la politique du logement et les difficultés rencontrées par ce secteur. La réduction de loyer de solidarité, destinée à compenser la baisse des APL dans le parc social, n'a pas manqué de produire ses effets. Je rappelle que, en imposant des baisses de loyer, le Gouvernement a voulu alors forcer, non sans brusquerie et avec un semblant de concertation, les organismes d'HLM à se restructurer. En contrepartie, le taux du livret A sera gelé à 0,75 % jusqu'en 2020, jusqu'en 2020, la dette des OLS sera allongée, des prêts haut de bilan et des prêts à taux fixes leur seront consentis, pour respectivement 2 milliards et 4 milliards d'euros, des avances de trésorerie leur seront accordées ... Les conséquences, je le disais, n'ont pas mis longtemps à se manifester, sous forme d'abandon ou de contraction de projets de construction de nouveaux logements sociaux et de réhabilitation. De son côté, l'Union sociale pour l'habitat, lors de son congrès annuel qui s'est tenu en octobre dernier, évoquait une baisse d'au moins 5 % des nouveaux logements prévus cette année. Pour ce qui concerne les permis de construire et les mises en chantier de logements neufs, les dernières données, celles du troisième trimestre de 2018, sont assez éloquentes. Depuis le début de l'année, la construction de logements neufs se contracte sérieusement 122 000 permis de construire, soit une baisse de 10,2 % par rapport à la même période en 2017, et 85 000 mises en chantier, soit une baisse de 7,9 %. Je voudrais également dire un mot sur le programme 135, « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

Ce programme devrait répondre à l'enjeu de créer un choc de l'offre dans les zones tendues, tout en assurant un développement équilibré des territoires. Or ce programme prévoit, avec 285 millions d'euros, inscrits en autorisations d'engagement et en une baisse de 7,4 % des crédits de paiement par rapport à l'année 2018. Je rappelle que ces crédits avaient déjà diminué de 22 % entre 2017 et 2018. Au titre des dépenses fiscales sur impôts d'État,

38 millions d'euros en 2018 et de zéro euro en 2019. Notre rapporteur spécial, dans son rapport d'information consacré à cette question, s'est d'ailleurs inquiété de la situation difficile du FNAP en raison du retrait massif de l'État du financement des aides à la pierre. Pourtant, le FNAP, au sein duquel l'État et des organismes d'HLM gèrent conjointement les fonds publics dédiés au développement et à l'amélioration du parc social, aurait besoin de territorialiser ces crédits en associant véritablement les élus locaux. C'est d'ailleurs le sens des recommandations qui vous ont été faites par Philippe Dallier,

bailleurs, à permettre au FNAP de financer des réhabilitations et pas seulement des constructions neuves, particulièrement dans les zones qui ont un parc ancien et dégradé, et enfin à généraliser les délégations des aides à la pierre aux collectivités locales.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, avec ce gouvernement, je dois le dire, lorsqu'il s'agit de politique de la ville, nous ne savons pas sur quel pied danser. 2017 avait été marquée par des discours ambitieux d'émancipation du Président de la République à Clichy-sous-Bois et Tourcoing, qui répondaient à la fronde massive des associations et des maires de toutes tendances traduite dans l'appel de Grigny, mais qui étaient dénués de réelles concrétisations budgétaires.

car, plus il y aura d'écoute, moins il y aura de « gilets jaunes » ! La politique d'émancipation en faveur des habitants des quartiers nécessite des moyens. L'émancipation passe par l'éducation, bien sûr, mais aussi par l'emploi. Dans nos quartiers prioritaires, le taux de chômage, je le rappelle, est de 27 %. En même temps, vous persévérez diaboliquement sur le chemin de la suppression d'un très grand nombre de contrats aidés. Le dispositif expérimental des emplois francs « nouvelle mouture » est en deçà des objectifs fixés. Au 1 septembre 2018, moins de 2 000 emplois francs auraient été conclus, quand 25 000 sont attendus à la fin de 2019. Remobiliser les préfets et s'appuyer davantage sur les missions locales est important, mais ce n'est pas suffisant. Dans ce domaine, nous croyons en « l'efficacité d'échelle ». Pourquoi donc ne pas étendre la liste des territoires éligibles à l'expérimentation au-delà des sept territoires actuels ? Concernant la rénovation urbaine, des inquiétudes demeurent. Si l'État semble confirmer son engagement pris au courant de l'année, nous nous retrouvons avec un financement du NPNRU de 185 millions d'euros en autorisations d'engagement et de seulement 25 millions d'euros en crédits de paiement. Nous comprenons l'argument qui consiste à expliquer que les projets de rénovation ne sont pas encore ficelés, mais nous avons perdu dix-huit mois. Ce délai, quand on connaît l'état d'insalubrité de nombreux logements et l'impact direct sur l'état de santé des habitants-

peut aussi être un facteur retardateur de la mise en place du NPNRU. Un des principaux acteurs de la politique de la ville, c'est le territoire, plus particulièrement la commune. Permettez-moi de le souligner, de ce côté-là, le compte n'y est pas. Arrêtons-nous un instant sur la dotation politique de la ville, la DPV. Vous annoncez l'avoir sanctuarisée à hauteur de 150 millions d'euros en 2019, mais vous élargissez le champ d'attribution de cette dotation. Cela signifie que l'enveloppe globale reste identique, mais que le nombre de villes concernées augmente. Ces villes toucheront donc, en moyenne, moins que l'année précédente. Examinons maintenant la dotation de solidarité urbaine. Si la péréquation horizontale n'augmente pas, la péréquation verticale augmente moins que toutes les autres années : cela représente 20 millions d'euros en moins par rapport au budget pour Chaque année, ces communes les plus pauvres de notre pays perdent des recettes si l'on tient notamment compte des abattements et exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous le savez, monsieur le ministre, que les communes soient rurales ou urbaines, ces dotations constituent pour elles la seule recette dynamique de leur budget. Cela ne peut plus continuer ainsi Il y a urgence sociale dans tous nos quartiers prioritaires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Face à l'ampleur des inégalités vécues par ces 5 millions de Françaises et de Français, la réponse républicaine doit être globale : sur l'éducation, sur l'emploi, sur le logement et sur le cadre de vie. Il y va de la survie de notre cohésion nationale. Car forcément funeste sera le destin d'un pays qui voit sa population partagée en deux nations : la nation des privilégiés, pour qui le champ des possibles est grand ouvert, et celle de ceux pour qui l'égalité des chances n'est qu'une chimère. Vous comprendrez que notre groupe s'abstiendra sur les crédits de la politique de la ville. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, jamais autant qu'aujourd'hui nous n'avons entendu parler de cohésion des territoires et, convenons-en, c'est plutôt une bonne chose. Aussi permettez-moi de rendre hommage à l'un de ceux qui ont permis qu'on en parle concrètement, l'élu d'un territoire ô combien symbolique et qui m'est cher de surcroît, qui n'a pas découvert la ruralité entre Bercy et l'Hôtel de Castries et qui n'a pas ménagé sa peine, dans des conditions particulièrement difficiles, pour défendre la cause de ces territoires que nous aimons tant. Je veux bien sûr parler de notre collègue Jacques Mézard,

Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Mettre en oeuvre une politique de l'aménagement du territoire en France, c'est disposer de l'expertise, des moyens et de l'autorité nécessaires pour faire vivre, au quotidien, la République des territoires. Or, depuis des décennies, force est de constater que nous avons assisté à un abandon en règle des territoires. Aujourd'hui, l'État doit impérativement avoir une vision stratégique. La France métropolitaine est, semble-t-il, entrée dans les moeurs : c'est un ressenti. Elle concentre déjà 75 % de la croissance : c'est une réalité ! Comme par hasard, on se rend compte maintenant que la métropolisation peut engendrer un phénomène ségrégatif : la belle affaire Bien sûr, il est nécessaire et urgent de promouvoir une politique spécifique pour les petites et moyennes villes, dont beaucoup ont de grandes difficultés, en particulier celles qui n'ont pas de noyau métropolitain. Bien sûr, il est nécessaire et urgent de venir en aide aux territoires laissés pour compte et qui s'enfoncent petit à petit dans le repli et la désertification. Ce n'est plus une fracture territoriale, c'est un abandon en rase campagne Alors, nous dit-on, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est certainement l'outil nécessaire pour que le territoire national ne fasse qu'un. Soit ! Le chef de l'État lui-même a indiqué, lors de la Conférence nationale des territoires, que le travail effectué fera en lien direct avec les régions et que l'agence apportera un appui en ingénierie publique aux territoires les plus périphériques, dans une logique de guichet unique et de simplification à destination des porteurs de projets et des élus. des élus. Selon ses termes, « ce que demande la ruralité, ça n'est pas l'aumône, ça n'est pas d'être compensé, c'est d'avoir les mêmes chances de réussir », et il défend une approche « différenciée » de l'État, qui « ne doit pas craindre de donner plus à ceux qui ont moins Il s'agit là du discours de façade, mais, « en même temps », qu'en est-il dans la réalité ? Depuis le fiasco de la Conférence nationale des territoires et de son double langage, la confiance n'est plus là là ! par exemple, des capacités financières ? Mes collègues rapporteurs Dominique Estrosi Sassone et Philippe Dallier l'ont dit précédemment, le compte n'y est pas. Le renversement du tropisme métropolitain, qui a prévalu lors de la funeste réforme territoriale, ne s'opérera pas avec de belles paroles Si je ne devais prendre qu'un seul exemple révélateur d'un aménagement du territoire chaotique et d'une cohésion des territoires à géométrie variable, je choisirais celui que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de mon département, l'Essonne. Dans la partie urbanisée, au nord du département, s'agissant d'un projet d'envergure nationale, le fameux plateau de Saclay, le Président de la République est venu sur place le 25 octobre 2017 nous parler, les yeux dans les yeux, en disant : « Je Je ne ferai rien qui pourra contrarier l'avenir du plateau de Saclay, ce coeur battant de la science française [ ...] Une grande partie des réponses aux défis contemporains vient d'ici [ ...] Il s'agit de gagner la bataille de l'intelligence [et] d'être à la pointe de l'excellence scientifique ». Parlons-en Quelques semaines après cette déclaration d'amour enflammée, le Premier ministre est venu, en service commandé, annoncer brutalement aux élus locaux, faute de crédits, un report en 2027 de l'avènement de la ligne 18 du Grand Paris Express, axe principal des transports en commun censés irriguer ce fameux plateau de Saclay. Dans le même temps, la partie périurbaine et rurale, plus au sud du département, le Gouvernement continue aveuglément d'intimer l'ordre aux élus locaux, sur les bases du sacro-saint article 55 de la loi SRU et à coups de constat de carence, de construire toujours plus de logements, alors même que les transports en commun sont déjà sursaturés le long des lignes C et D du RER, dont la réputation n'est plus à faire Est-il besoin de rappeler ici la mémoire des sept morts lors du drame de Brétigny-sur-Orge, le 12 juillet 2013, par manque d'entretien du réseau ? Voilà quelle est la réalité de la cohésion des territoires, au moins dans le département de l'Essonne. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre, nous n'avons pas besoin d'usine à gaz administrative, pas plus que de discours lénifiants. Nous avons besoin de confiance et d'actes concrets ! La parole est

Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous à l'occasion de l'examen de la mission « Cohésion des territoires ». Je voudrais d'ailleurs vous remercier à la fois de la qualité et de la précision des différents échanges que nous avons pu avoir, soit en amont de cette

avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant près d'un an et demi. Nous avons mené de grands combats, lancé de nombreuses initiatives et partagé cet objectif que nous avions déjà en commun lors de la campagne présidentielle, à savoir la lutte sans relâche contre les fractures territoriales encore

les événements qui se déroulent actuellement dans notre pays- le fameux mouvement des « gilets jaunes » -sont le reflet de ces fractures territoriales qui perdurent dans notre pays. Au-delà du ras-le-bol fiscal, pour

pour ne jamais faire d'amalgame avec une seule ruralité, qui ne fait pas sens, en tout cas pas à mes yeux. Ces fractures alimentent le sentiment de relégation, et parfois d'abandon. Tout l'enjeu du ministère

Je voudrais d'abord insister sur ce bras armé de la politique de l'aménagement du territoire qu'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, que le Président de la République avait annoncée et qui va être créée. Je voudrais saluer votre implication à toutes et tous

Je suis convaincu que vous êtes nombreux à partager sur ces travées un autre constat que nous faisons : nos politiques publiques en matière d'aménagement, de logement ou de politique de la ville doivent être

du programme « Action coeur de ville », qui vise à rénover l'habitat, mais aussi à redynamiser l'économie ou, à tout le moins, le tissu commercial de villes dites de « taille moyenne »- je pense à des sous-préfectures ou à des préfectures de petite taille -, lesquelles ont peut-être été trop longtemps les oubliées des politiques d'aménagement du territoire et du logement.

Autrement dit, les acquisitions de logements anciens faisant l'objet d'au moins 25 % de travaux de réhabilitation pourront donner lieu à

conclure à cette date. Deux sujets seront étudiés en toute transparence et les parlementaires seront associés aux travaux. Le premier porte sur la situation financière des bailleurs et les perspectives à court et à moyen terme ; le second, sur les bilans chiffrés de la RLS, de la hausse de la TVA

le jour même, et y suis retourné toute la journée, hier, pour accompagner les Marseillaises et Marseillais et mettre en avant des mesures fortes à la fois d'accompagnement, mais aussi de suivi

menés actuellement sous l'égide du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Bien évidemment, quand on parle d'insalubrité, il faut évoquer la question de la rénovation des bâtiments.

de ce que nous pouvons faire pour accompagner toutes celles et tous ceux qui sont dans ces situations de détresse. Cela passe notamment par les financements supplémentaires que nous avons consacrés aux maraudes, mais également par le plan Logement d'abord,

L'objectif assumé du Gouvernement est d'inciter le secteur du logement social à s'autonomiser, en finançant ses nouveaux projets par la vente d'une partie de son patrimoine. Le désengagement complet de l'État des aides à la pierre est inacceptable et rompt l'équilibre qui a prévalu à la création du FNAP en 2016 : une parité de financement entre l'État et les bailleurs, et une gouvernance équilibrée organisée autour de l'État, des collectivités territoriales et des bailleurs.

Cet amendement tend à inscrire la contribution de l'État au financement du FNAP à hauteur de 200 millions d'euros ; il s'agit d'un enjeu de solidarité nationale. Au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre du plan Logement d'abord, qui doit accélérer la production de logements sociaux et très sociaux, il paraît nécessaire que les crédits

des financeurs- l'État, les bailleurs sociaux -, pour que la programmation tienne bien compte des besoins des territoires et de leurs capacités à agir.

Tout cela ne fonctionne que si les fonds propres des organismes permettent à ceux-ci d'agir. C'est une espèce de jeu de cubes : quand il manque quelque chose dans le dispositif, tout s'écroule. Donc, effectivement, le prélèvement et la RLS fragilisent les capacités d'investissement des organismes.

sociaux n'ont plus les moyens d'assurer leur propre financement. Donc on va se trouver avec un résultat exactement inverse de ce que l'on cherche : promouvoir la construction de logements sociaux et très sociaux.

Le Gouvernement affirme que sa politique redonne du pouvoir d'achat aux ménages et protège mieux les familles modestes, mais, au regard de cette volonté affichée, il nous paraît nécessaire que les crédits du programme 109 soient majorés en conséquence par le Gouvernement, sans faire supporter cet effort au programme 177 de la mission. Quel est l'avis

dirions que vous recalez l'effort en le positionnant de sorte que les choses soient plus simples, plus immédiates, plus fluides et plus justes ; soit, mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous faites de l'économie budgétaire et, pendant le même temps- bonjour la justice sociale, parce que les bénéficiaires de l'APL ne sont tout de même pas les plus riches du pays

une proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, ou ANCT. Le présent amendement vise à donner à cette future agence les moyens de ses missions et de ses ambitions, puisqu'elle sera un acteur central au croisement de tous les tous les opérateurs- ANAH, ANRU, CEREMA, ADEME -qui fournissent aux collectivités territoriales des moyens d'ingénierie en matière d'urbanisme, de construction, de mise aux normes ou encore de développement durable. le contexte budgétaire contraint dans lequel évolue le programme 112, « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », marqué par plusieurs années d'affaiblissement en loi de finances- baisse en crédits de paiement, par rapport à 2018 -ne garantit pour l'instant pas à la future ANCT la robustesse financière dont elle aura besoin pour assurer correctement ses missions. C'est d'autant plus vrai que le Commissariat général à l'égalité fait l'objet dans le PLF pour 2019 de plusieurs suppressions de poste. Si nous voulons que l'agence soit structurante pour le maintien des services publics, la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, la transition écologique, ou encore l'accès aux soins et au numérique, il est indispensable de reconsidérer largement le niveau de ses crédits. C'est d'autant plus nécessaire- cette crainte a déjà été exprimée par nombre d'entre vous -qu'il nous faut également remédier au risque d'une trop grande asymétrie entre l'action urbaine de l'agence et son action rurale, eu égard à l'importance du programme 147, « Politique de la ville », par rapport au programme 112, dont l'ANCT a vocation à devenir le pilote, en remplacement du Commissariat général

112, dans la perspective de la mise en oeuvre opérationnelle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Jusque-là, on est d'accord ; mais comment financer ces 80 millions d'euros ? Cet amendement tend à réduire, à hauteur de 65 millions d'euros, le programme 135

Merci

Monsieur le ministre, en vous écoutant pendant les vingt minutes où vous avez répondu aux différents orateurs, j'ai été un peu étonné : à aucun moment vous n'avez vraiment évoqué les nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus du logement, alors que presque tous nos collègues en ont

L'APL accession a vocation à soutenir des ménages aux revenus modestes dans les zones détendues, particulièrement dans les centres-bourgs, et parfois dans des zones où il n'y a pas d'offre locative adaptée pour ces familles. Dans nombre de cas, le projet d'acquisition n'aurait pas pu être possible sans le soutien de l'APL accession, qui intervient comme un réel déclencheur. Cette aide a souvent été nécessaire pour conforter un prêt aidé ; pour les ménages du premier quartile, elle permet de réduire d'un quart les mensualités de remboursement. Sa suppression, voulue par le Gouvernement, est bien contre-productive : elle a pour effet de bloquer la mobilité des ménages les plus modestes. Elle n'est pas non plus cohérente avec les objectifs du Président de la République, pour vendre 40 000 logements sociaux à leurs locataires, il faudra accompagner les ménages, qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens d'acheter. L'APL accession est de nature à accroître la mobilité dans le parc social et à faciliter la vente de logements HLM à leurs locataires. plus, en soutenant les ménages, on soutient aussi l'activité du bâtiment, alors que, comme vous le savez, monsieur le ministre, les chiffres de la construction sont en baisse. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter les crédits du programme 109 de 50 millions d'euros, qui correspondent au coût estimé du dispositif pour un an.

», n'ont plus d'outils pour l'accession sociale à la propriété. Il n'y a plus d'aides publiques de l'État dans ces territoires ! Or, pour une partie des familles concernées, l'accession est une forme de promotion

une aide de l'État versée aux communes qui font partie d'une zone tendue et mènent un effort particulier en matière de construction. Cette aide, mise en place en 2015, répondait à une demande forte de l'ensemble des élus locaux. En 2015, 472 communes en ont bénéficié, pour un montant global de 35 millions d'euros.

Le Gouvernement a supprimé cette aide votée par le Parlement, sans aucune évaluation. Soutenir les communes qui font les efforts nécessaires pour améliorer l'accès au logement de nos concitoyens nous paraît pourtant essentiel. essentiel. Nous proposons donc de rétablir pour 2019 les crédits de l'aide aux maires bâtisseurs à hauteur de 45 millions d'euros. Au regard de la volonté du Président de la République de créer un choc de l'offre, il paraît nécessaire que les crédits de l'aide aux maires bâtisseurs soient abondés par le Gouvernement sans faire supporter cet effort par un autre programme de la mission.

Sans la moindre consultation préalable, le Gouvernement a publié le 2 mai 2018 un arrêté national fixant des tarifs plafonds par groupe homogène d'activité et de mission. De telles réductions budgétaires impactent lourdement les CHRS, menacent la pérennité de certains d'entre eux et se traduiront rapidement par une baisse de la qualité des services et par un accompagnement social Ces centres jouent pourtant un rôle majeur dans l'accompagnement, l'hébergement et la réinsertion sociale de personnes en situation de grande difficulté : jeunes en errance, femmes victimes de violence, personnes précaires atteintes de troubles psychiques ou encore familles en situation de très grande précarité. cet amendement, nous proposons de maintenir pour 2019 les crédits alloués aux CHRS au niveau de ceux de l'année 2018, soit une augmentation de 13,4 millions d'euros. Au regard des engagements pris par le Président de la République dans le cadre du plan Logement d'abord, qui nécessite un effort accru en faveur de l'accompagnement social,

demande le retrait

Cet amendement vise à abonder les crédits du programme 112, « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », consacrés à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services, Cette aide directe à l'investissement pour les entreprises porteuses de projets innovants, versée en contrepartie de la création ou du maintien d'emplois, paraît actuellement sous-dotée dans le présent PLF, alors que tous les indicateurs montrent qu'il s'agit d'un dispositif efficace. efficace. Alors même que les besoins de la PAT sont estimés dans une fourchette comprise entre 30 millions et 35 millions d'euros, le PLF 2019 lui consacre à peine 10 millions d'euros, soit trois fois moins que ce qui lui serait nécessaire pour le ministre, mes chers collègues, vous connaissez comme moi l'impérieuse nécessité de préserver des bassins d'emploi dans les territoires, en particulier dans ceux qui sont les plus en difficulté. 75 % des projets primés par la PAT sur la période 2010-2017 étaient situés dans des territoires à forts enjeux : communes rurales, villes moyennes, quartiers de la politique de la ville ou zones de revitalisation rurale. En ce sens, la PAT est donc l'un des outils les plus efficaces parmi ceux qui sont mis à la disposition des acteurs économiques locaux, en complément du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT. Entre 2014 et 2017, la PAT a en effet accompagné la création ou le maintien de plus de 39 000 emplois. Pour un euro de PAT distribué, 26 euros étaient investis en 2018 par les entreprises bénéficiaires, contre 42 euros attendus en 2020. En conséquence, nous proposons ce rééquilibrage cohérent avec l'efficience et les besoins réels de la PAT. Très bien

En prévoyant que les logements seront « évolutifs » à l'issue de « travaux simples », le Gouvernement fait peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte d'engager des travaux d'adaptabilité.

Au regard de l'engagement du Président de la République de faire du handicap une priorité de son quinquennat- une de plus ! -, il paraît nécessaire que les crédits de l'ANAH soient abondés en conséquence par le Gouvernement, sans faire supporter cet effort au programme 109 de la mission.

dire un mot sur le financement de l'ANAH. Sur ce sujet, je n'aime pas parler en chiffres. Je comprends bien que le Gouvernement se fixe toujours des objectifs. Vous nous dites : on va passer de 50 000 à 75 000, mais je vous renvoie aux conclusions

Pendant plus de vingt ans, malgré les interdictions d'utilisation, l'État a tout de même continué de délivrer des agréments pour un produit que l'on découvre aujourd'hui comme étant le pire de ce que l'on a pu produire dans le domaine phytosanitaire.

Le Président de la République s'est rendu à la Martinique et à la Guadeloupe- les deux départements touchés -voilà quelques semaines. Il a assuré le scandale d'État, il a assumé le scandale d'État.

Aujourd'hui, des produits continuent d'être vendus en bord de route, sur des marchés parallèles, etc., sans que l'État ait les moyens de pouvoir contrôler s'ils sont propres ou impropres à la consommation.

en faveur de ce plan, soit le même niveau que l'année passée. Elle a également rappelé les engagements du Président de la République pour renforcer les crédits, et c'est nécessaire. Nous allons voir quel sera l'avis du Gouvernement

; cet engagement sera tenu la gestion et non pas un crédit budgétaire additionnel d'un programme.

une volonté écrite, une volonté dite, une volonté annoncée, une volonté proclamée, qui n'était pas de l'incantation, parce que le Président y a mis les formes, regrettant même

prendra donc la forme d'un amendement d'appel. Le projet annuel de performance de la mission « Cohésion des territoires » précise que l'action n° 03, Lutte contre l'habitat indigne, du programme 135 financera à hauteur de 17 millions d'euros un nouveau dispositif d'aide aux travaux. Cet amendement d'appel est destiné à obtenir des précisions de la part du Gouvernement sur cette subvention. Quelle part sera réellement affectée à la réhabilitation des logements outre-mer et selon quelles modalités ? Quel

mais, monsieur le ministre,